portant sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative, notre collègue Véronique Guillotin a été notée comme ayant voté pour alors qu'elle souhaitait s'abstenir.

un rappel au règlement. La liberté de parole des parlementaires dans l'exercice de leur mandat est un principe fondamental reconnu par tous depuis la Révolution française. Au nom de la démocratie, certains soi-disant bien-pensants voudraient pourtant imposer une dictature de la pensée unique. Plus précisément, ils n'acceptent la démocratie que si l'on pense comme eux. Or je rappelle que l'article 26 de la Constitution garantit la liberté d'expression au sein du Parlement. De plus, la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2018 indique : « Toutefois, le règlement du Sénat ne saurait avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la liberté d'opinion et de vote des sénateurs. » Le 29 octobre dernier, les débats du Sénat concernaient le port du voile islamique par les personnes accompagnant les sorties scolaires des enfants. suite de mon intervention, M. Assouline, vice-président socialiste du Sénat, a saisi le bureau du Sénat et réclamé des mesures à mon encontre afin que je ne puisse plus m'exprimer librement. Non seulement il n'y est pas parvenu, mais je maintiens tout ce que j'ai dit : je ne retire absolument rien, ni à mon intervention du 29 octobre dernier ni à celle du 13 octobre 2015 sur le terrorisme.

Il s'agit là d'une diffamation pure et simple : le des débats du 29 octobre dernier prouve que je n'ai absolument jamais fait allusion ni à une race ni à un problème racial. Ce n'est pas la première fois que M. Assouline, agissant en tant que vice-président socialiste ou en tant que président de séance du Sénat, m'agresse avec une totale mauvaise foi. C'est inacceptable et je souhaite que, à l'avenir, le Sénat veille à faire respecter la liberté de parole de chacun dans l'hémicycle

examinions la semaine dernière le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et que les débats nous ont une fois de plus montré combien il était difficile de parvenir à l'équilibre des comptes sociaux, cette proposition de loi vise à instituer un nouvel outil afin de renforcer le caractère protecteur de notre système de santé. Nous abordons un sujet complexe complexe : de nombreuses études, de multiples rapports établis par différentes administrations et missions parlementaires donnent des estimations très variées sur l'ampleur de la fraude à la carte Vitale. Les chiffres avancés varient de 1 million d'euros à plusieurs centaines de millions d'euros par an. an. Sommes-nous vraiment capables d'estimer l'ampleur de la fraude à l'assurance maladie et, tout spécialement, de la fraude aux cartes Vitale ? Quoi qu'il en soit, de nombreux indicateurs laissent à penser que cette fraude est importante. À titre d'exemple- il ne s'agit pas d'une simple anecdote -, il est possible d'acheter une carte Vitale au marché noir pour environ 50 euros. Ce n'est pas cher ! Derrière cette fraude se dessine une réalité tangible qui, si elle n'écornait pas autant le pacte républicain, pourrait prêter à sourire.

comment imaginer que le nombre de cartes Vitale actives dépasse le nombre de bénéficiaires effectivement couverts, et ce dans de telles proportions ? Les estimations varient entre 2 et 5 millions. Comment accepter que des personnes utilisent régulièrement une carte Vitale attribuée à une autre ? Comment comprendre que l'Insee recense près de 3 millions de centenaires en France ? Ces différentes incohérences exigent des réponses, car elles causent un préjudice financier non négligeable à notre système de santé. Au regard du poids qu'occupe l'assurance maladie dans les dépenses publiques, elles-mêmes déjà considérablement sous tension,

Depuis 2005, l'assurance maladie a mis un terme à 2,4 milliards d'euros de fraudes ou d'activités fautives. Si les estimations sont très difficiles à établir en la matière, les occasions de fraude sont, en tous les cas, nombreuses.

: la carte Vitale biométrique serait un instrument de lutte contre la fraude à la carte Vitale classique, grâce à l'image numérique des empreintes digitales du titulaire qu'elle contiendrait.

Aussi, quand bien même son coût pour les dépenses publiques serait modique, la fraude n'est pas, et ne doit pas être, une variable d'ajustement. Il n'est en aucun cas question de stigmatiser ceux d'entre nous qui sont les plus défavorisés ou de flécher telle ou telle partie de la population. Il s'agit, en revanche, de préserver un principe : l'intérêt général, en vertu duquel les droits accordés au citoyen impliquent en contrepartie des devoirs, au premier rang desquels celui de ne pas frauder. Ne pas chercher à préserver ce principe, c'est mettre en danger l'intérêt collectif et la pérennité de notre système de soins. Lorsque nous échangeons avec les professionnels de santé, nous constatons que beaucoup d'entre eux sont démunis face aux usurpations d'identité au moyen de la carte Vitale. rôle n'est d'ailleurs pas d'effectuer des contrôles. La mise en place d'une carte Vitale biométrique devrait leur permettre de se protéger face à ce type de situations frauduleuses.

Ainsi, la commission a adopté une nouvelle rédaction de l'article 1, qui prévoit la mise en place d'une carte Vitale biométrique expérimentale, avec un enrôlement obligatoire des bénéficiaires. Cette expérimentation, qui pourra porter sur quelques caisses de sécurité sociale réparties sur l'ensemble du territoire national, permettra non seulement de tester la faisabilité technique et financière du déploiement de cette carte Vitale biométrique,

Dans tous les cas, cette expérimentation sera l'occasion d'avoir, définitivement, une idée plus précise de l'ampleur de la fraude à la carte Vitale. Les élus du groupe Les Républicains souhaitent donc l'adoption de ce texte, tel qu'il a été modifié par la commission des affaires sociales. Très bien

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de nos collègues Philippe Mouiller, Bruno Retailleau et Alain Milon tendant à instituer une carte Vitale biométrique. Comme il s'agit d'un sujet sensible, susceptible de déclencher promptement des procès d'intention, je tiens à rappeler que les débats au sein de la commission des affaires sociales ont permis l'émergence d'une solution approuvée, sinon par tous les groupes, par la majorité d'entre eux. Ensemble, nous nous sommes entendus pour réaffirmer la nécessité, dans des temps critiques où les fondements de notre pacte républicain sont plus fragilisés que jamais, de raffermir le juste versement des droits à travers la sécurisation des titres qui y donnent accès. Ensemble, nous sommes convenus qu'il était vain et stérile d'opposer les fraudes entre elles, qu'elles soient sociales ou fiscales, alors qu'elles procèdent toutes du même fléau. Certes, les moyens mis en oeuvre pour lutter contre la fraude doivent rester proportionnés au préjudice financier qu'ils combattent mais tout acte frauduleux, quelle que soit son ampleur, porte une atteinte intolérable à cette juste attribution des droits. Il convient de rappeler que la carte Vitale ouvre droit uniquement à des prestations d'assurance maladie, non aux autres prestations sociales, qui participent elles aussi de la fraude sociale. étant, son usage abusif ne fait pas qu'obérer le budget de la sécurité sociale : il touche la solidarité nationale au coeur tout en entretenant doutes et suspicions. le préjudice financier lié à la fraude à la carte Vitale n'est peut-être pas le plus significatif, mais des incertitudes demeurent quant à son chiffrage. En outre, cette fraude est l'une de celles dont l'occurrence est la plus fréquente ; et c'est celle qui porte le plus visiblement atteinte à la solidarité nationale. C'est donc à un dommage aussi financier que symbolique que le présent texte entend s'attaquer. La proposition de loi initiale défendait une idée ambitieuse : substituer des cartes Vitale biométriques à l'ensemble des cartes Vitale existantes.

Compte tenu de la sensibilité de la question biométrique, la commission n'a pas souhaité que l'attribution généralisée de cette nouvelle carte Vitale donne lieu à la constitution d'une base de données où seraient consignées les empreintes digitales numérisées de tous nos concitoyens. et des libertés (CNIL) n'a pas manqué de nous le rappeler. Par ailleurs, l'attribution d'une carte Vitale biométrique doit tenir compte des chantiers déjà lancés par le Gouvernement en la matière.

fait intervenir l'élément biométrique, mais uniquement lors de l'enrôlement : le bénéficiaire est alors invité, et non contraint, à une identification biométrique lors de l'attribution de la carte, dont l'usage sera par la suite simplement conditionné à la présentation de son téléphone portable. est intéressante, mais elle ne garantit pas vraiment la stricte identification. Les téléphones se prêtent certes moins facilement que les cartes Vitale actuelles. Toutefois, ils circuleront sans aucun mal dans les cercles intrafamiliaux, qui sont précisément ceux où la fraude est la plus pratiquée. De plus, l'attribution fondée sur le volontariat et la distribution limitée aux seuls bénéficiaires équipés d'un support mobile nous feraient, sans aucun doute possible, manquer la cible que notre proposition de loi a identifiée comme devant être visée par la biométrie, à savoir les fraudeurs. Pour autant, nous n'avons pas souhaité, par réalisme, que notre proposition « écrase » l'expérimentation en cours. La commission a même considéré que les deux dispositifs pourraient être utilement déployés de concert : l'on pourrait ainsi livrer, d'ici un an, leurs résultats comparés. C'est le sens de la modification que nous avons apportée à l'article 1, en substituant à la carte Vitale biométrique généralisée une carte Vitale biométrique expérimentale, testée dans un nombre limité de territoires.

afin que soient bel et bien anéantis les risques de fraude en obtention des droits. Un enrôlement total permettra de mettre un terme au problème persistant des cartes surnuméraires, dénoncé dans leur rapport par nos collègues Mmes Nathalie Goulet et Carole Grandjean. collègues, tel est le sens des modifications que nous avons apportées à cette proposition de loi. Nous en avons conservé le principe et n'en avons modifié les contours, avec l'accord de ses auteurs, que pour permettre son effectivité ! Bravo ! La parole

la fraude détectée par les organismes de sécurité sociale s'est élevée à 1,2 milliard d'euros, ce qui correspond à une hausse de plus de 40 % en quatre ans. La proposition de loi dont nous allons débattre cette après-midi porte sur le sujet particulier de la fraude à l'usage de la carte Vitale. Vous le savez, la carte Vitale permet d'établir des feuilles de soins électroniques, documents servant de base au remboursement ; mais ce n'est pas sa seule fonction au regard de la situation des assurés. sert aussi à gérer leurs droits, qui sont historiquement inscrits dans la carte et accessibles directement, en cohérence avec les droits ouverts et contrôlés par les caisses d'assurance maladie. La fraude à l'usage de la carte Vitale repose sur une usurpation de carte : une personne sans droits utilise la carte d'une personne ayant des droits ; une autre utilise celle d'une personne couverte à 100 % alors qu'elle-même n'a que des droits à la couverture de base.

Je tiens à revenir sur les nombreuses mesures prises depuis 2004 pour réduire les risques liés à la délivrance de la carte et sécuriser tout à la fois notre système d'émission des cartes et les facturations facturations : la création d'une liste d'opposition des cartes Vitale, qui permet de bloquer l'utilisation des cartes mises en opposition ; l'ajout de la photographie en couleur de l'assuré, tant sur le support de la carte que dans le composant électronique la mise en place d'un portail interrégimes, qui permet d'éviter l'émission d'une nouvelle carte si l'ancienne n'a pas été restituée ou invalidée ; enfin, la mise en fin de vie des cartes Vitale dont les titulaires n'ont plus de droits, sont décédés ou radiés.

Ces compléments seraient ensuite utilisés par les professionnels de santé pour vérifier la bonne correspondance entre le titulaire de la carte et la personne qui l'utilise. La commission a modifié cette proposition de loi, qui privilégie désormais la voie de l'expérimentation.

L'utilisation des empreintes induit des coûts et des délais de mise en oeuvre importants pour le recueil des données biométriques, le contrôle par les professionnels de santé et l'adaptation du système de gestion des cartes Vitale.

Pour exercer un contrôle biométrique, il serait aussi nécessaire que les professionnels de santé soient équipés d'un matériel permettant de relever les empreintes du patient. Ce processus aurait

leurs missions. Au-delà de la polémique que ce changement pourrait créer avec les professionnels utilisant la carte Vitale au quotidien, un financement de ces matériels par l'assurance maladie serait demandé. Enfin, les contraintes de sécurité afférentes à l'utilisation des données biométriques par des traitements automatiques induisent une complexité technique. La mise en place de cette nouvelle carte serait de nature à augmenter de façon substantielle le prix unitaire de la carte Vitale et, plus généralement, le coût global de gestion des cartes.

Ce dispositif présente une forte valeur ajoutée pour lutter contre la fraude : il permettra une mise à jour des droits en temps réel, ce qui ne serait pas le cas avec la carte Vitale biométrique proposée. expérimentation est régie par le décret du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une e-carte d'assurance maladie. Actuellement menée dans deux départements, le Rhône et les Alpes-Maritimes, Alpes-Maritimes, elle est nécessaire pour évaluer et, si besoin, consolider l'ensemble du processus afin de sécuriser la délivrance de cette application, qui, dans un premier temps, cohabitera avec la carte physique.

Madame la présidente, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, je tiens à vous féliciter d'avoir repris à votre compte l'engagement présidentiel n° 71 de Marine Le Pen, ... Eh oui ! ... qui vise à instaurer une carte Vitale biométrique pour lutter contre la fraude documentaire aux prestations sociales. Dans ce même engagement, Marine Le Pen proposait de réaliser des économies supplémentaires en supprimant l'aide médicale d'État (AME), scandaleusement réservée aux clandestins, et de baisser le prix des médicaments coûteux l'augmentation de la proportion de génériques. Mais ça, ce sera pour 2022 Votre proposition de loi n'est qu'un pas, un premier et tout petit pas ; or, dans ce domaine comme dans tant d'autres, il y a urgence à changer radicalement de cap, car les chiffres issus du rapport d'information de notre collègue sénatrice de l'Orne ont de quoi donner le vertige. Le coût des fraudes aux prestations sociales

Avec plus de 2 200 milliards d'euros de dette, nous continuons de donner un « pognon de dingue », un « pognon » que nous n'avons pourtant pas ! Au total, 5 millions de cartes Vitale sont actives frauduleusement. Selon le répertoire national d'identification des personnes physiques, notre pays plus de 3 millions de centenaires, dont la plupart touchent des prestations, alors qu'ils ne seraient que 250 000 selon l'Insee. Pour couronner le tout, les organismes sociaux refusent, malgré de nombreuses relances, de communiquer à des parlementaires accrédités par le Gouvernement le nombre exact de personnes qui perçoivent des prestations. Pourquoi une telle omerta, alors qu'il s'agit de l'argent public ? Les Français ont le droit de savoir à qui bénéficie la solidarité nationale, qui est puisée- je vous le rappelle -dans leurs impôts Le secret imposé ne dissimulerait-il pas en réalité, au mieux l'incurie des services, au pire une fraude encore plus colossale que celle qui est annoncée ? Plutôt que de combattre cette fraude, qui ressemble au plus grand et au plus long braquage de l'histoire, l'on préfère, et ce sous tous les gouvernements, augmenter la pression fiscale et baisser le niveau de protection de ceux qui respectent la loi : c'est la double peine appliquée à ceux qui ne fraudent pas Il faut donc se doter, et urgemment, de moyens qui permettent de rétablir la justice sociale. Il faut désormais miser sur l'automatisation et la centralisation des données, ainsi que sur le recoupement des fichiers ; mais il faudra également multiplier les contrôles. Pour cela, la création d'une carte Vitale biométrique fusionnée avec le titre d'identité aurait constitué un changement radical, et une réforme bien plus aboutie, pour mettre un terme à cette gigantesque arnaque. Enfin, à l'heure des big data et du stockage d'informations, il convient d'avoir des fichiers fonctionnels et de fournir des chiffres fiables, pouvant être exploités efficacement en vue de redresser les comptes publics, et ce en toute transparence pour les Français. C'est ici une réforme structurelle qu'il faut avoir le courage de mener : elle va de pair avec la lutte contre l'immigration et la lutte contre une fiscalité abusive. Ce sont là trois points qui font la raison financière et qui ne pourraient que nous éclairer, mes chers collègues. Je voterai néanmoins ce texte et je veillerai à ce que, à l'avenir, une réforme plus aboutie

de pertes fiscales aux États du monde entier. Cette fraude remet en cause le principe d'égalité de tous les citoyens face à l'impôt. Elle ampute les recettes publiques de centaines de milliards d'euros, qui auraient dû financer l'éducation ou la santé. La fraude a de multiples facettes et nous regrettons que la majorité sénatoriale fasse le choix de s'attaquer en priorité à la fraude aux prestations sociales, qui est pourtant très loin d'être la plus importante.

? Même si nous n'acceptons pas les comportements frauduleux, il est légitime de s'interroger sur la pertinence et les raisons de ce choix. D'autres types de fraudes, qui pourraient rapporter bien davantage si elles étaient combattues,

dont le coût est évalué, en France, à environ 80 milliards d'euros par le syndicat Solidaires Finances publiques. Mes chers collègues, votre objectif est-il réellement de lutter contre la fraude,

Alors que les politiques de santé des dernières années cherchent à réduire le temps administratif des médecins, voulez-vous vraiment leur demander de contrôler les informations de la carte Vitale ? Si vous entendez vous attaquer à la fraude à la sécurité sociale, vous devriez également regarder du côté de certains professionnels de santé. santé. Selon les chiffres de 2018 de l'assurance maladie, 47 % de la fraude provient des offreurs de soins et de services, 30 % des établissements, et seulement 23 % des assurés sociaux. Il est dommage que vous ne prévoyiez aucune sanction à leur encontre. Contrairement à ce que laisse penser ce texte, la carte Vitale est seulement une carte à puce permettant aux professionnels de santé de connaître les droits du titulaire ou de ses ayants droit. Ce n'est pas une carte de paiement,

nous gardons de faire un amalgame entre le Rassemblement national et Les Républicains à propos de cette proposition de loi, nous regrettons que vous vous engagiez sur le terrain de l'extrême droite en stigmatisant les assurés sociaux et les personnes étrangères. Les futures échéances électorales ne sauraient justifier le renforcement d'idées populistes et xénophobes, bien trop présentes actuellement dans notre pays. La majorité sénatoriale aurait été mieux inspirée de s'en prendre à d'autres types de fraudes, je le répète, ou d'agir contre le non-recours aux prestations. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe CRCE votera contre cette proposition de loi. La

L'objectif de cette proposition est louable : il s'agit de lutter contre la fraude à l'assurance maladie en vérifiant l'identité de l'utilisateur d'une carte Vitale par un contrôle de ses empreintes digitales.

de lecture d'empreintes digitales. Par ailleurs, le rapporteur général de la commission des affaires sociales nous a fait part en réunion du projet du Gouvernement de mettre en place des cartes Vitale dématérialisées. Ces e-cartes

la fin mai 2020. Il fonctionne grâce à une application téléchargeable, permettant l'identification et l'authentification numérique des assurés, ainsi que le remboursement des actes et prestations. Cette carte Vitale 2.0 est délivrée sur demande pour une durée de douze mois. La généralisation du dispositif, après son

de limiter les risques de fraude, dans la mesure où il repose, pour le moment, sur le volontariat et où il n'aurait pas vocation à remplacer complètement la carte Vitale physique, laquelle resterait fonctionnelle. Aussi propose-t-il une solution de remplacement : le déploiement, à titre expérimental, d'une carte Vitale biométrique dans quelques caisses de sécurité sociale,

de demander à chaque assuré d'envoyer chaque année à sa caisse de sécurité sociale un justificatif de domicile, ainsi que la photocopie d'une pièce d'identité. Il faudrait également veiller à désactiver les cartes en cas de décès ou de manquement aux obligations de contrôle. Selon le Selon le rapport de la sénatrice Nathalie Goulet et de la députée Carole Grandjean, le coût de la fraude à la sécurité sociale est difficile à évaluer, mais il pourrait s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros par an. Le montant de la fraude aux faux numéros de sécurité sociale atteindrait, lui, entre 117 et 138 138 millions d'euros par an. D'un autre côté, le non-recours aux droits touche 28 % des assurés, qui ne bénéficient pas des prestations et des remboursements auxquels ils auraient droit. Nous devons agir agir pour plus de justice sociale, en limitant le risque de fraude, tout en favorisant le recours aux droits des assurés. Je serai attentif aux amendements déposés par la sénatrice Nathalie Goulet à ce sujet lors de l'examen en Ses propositions visent, notamment, à mettre en cohérence la durée de validité de la carte Vitale avec celle des droits de l'assuré. Il s'agit de renforcer le socle de la solidarité nationale, qui repose avant tout sur la juste utilisation des droits de chacun.

à l'enregistrement obligatoire, gratuit et public des naissances, ainsi qu'à la reconnaissance juridique des enfants sans identité,

Nous sommes ainsi passés d'une mesure d'ampleur visant à remplacer, pour l'ensemble des bénéficiaires de prestations d'assurance maladie, la carte Vitale actuelle par une carte Vitale biométrique à une expérimentation localisée. Votre rapport est sans appel, madame la rapporteure, ce que masquent mal les circonvolutions de forme auxquelles vous vous livrez pour ne pas fermement rejeter cette proposition. Ainsi, vous écrivez très justement que « la fraude à la carte Vitale ne représente qu'un montant faiblement significatif

représente moins de 5 % du montant total des fraudes aux prestations d'assurance maladie détectées. Plus précisément, la part de la fraude en obtention des droits strictement liée à l'usurpation de la carte Vitale a donné lieu au recouvrement d'un million d'euros en 2018, c'est-à-dire 0,5 % de la fraude à l'assurance maladie.

On aimerait pouvoir bénéficier d'estimations aussi précises concernant la fraude fiscale, mais l'observatoire promis il y a plus d'un an par le Gouvernement peine toujours à voir le jour. Qu'à cela ne tienne, Nathalie Goulet et Carole Grandjean, dans leur rapport dédié, placent également la focale sur la fraude sociale, notamment sur la fraude aux cartes Vitale, en expliquant sur les plateaux- sans chiffres à l'appui -que celle-ci est sous-estimée et représenterait des milliards d'euros.

par Nicolas Sarkozy en 2012, ce sont aujourd'hui les libéraux de tous bords qui tentent, une fois de plus, de surfer sur la vague de l'incurie de nos organismes de sécurité sociale. Ces organismes, ainsi que l'Insee, ont d'ailleurs fortement réagi pour rétablir la vérité sur le nombre de cartes Vitale

Ainsi, la cause principale de ce surnombre viendrait du simple usage et non d'une fraude organisée à grande échelle. Rappelons que, lors du lancement de la carte en 1998, un changement de situation ou de région entraînait l'édition d'une nouvelle carte sans restitution obligatoire de l'ancienne.

Un lent travail de désactivation des cartes Vitale en doublon a depuis lors été entrepris par les organismes compétents et des mesures antifraudes ont été mises en oeuvre. Au-delà de ces réticences, sur le fond, si nous devions prendre au sérieux la proposition initiale, la mise en place d'une carte Vitale biométrique aurait un coût prohibitif, évalué à près d'un milliard d'euros. Une telle disproportion nous invite, mes chers collègues, à envisager d'autres voies plus efficientes de modernisation de notre dispositif de lutte contre la fraude.

Autre problème d'ordre pratique : si seul le détenteur de la carte est en capacité de faire valoir ses droits, de la personne se rendant à la pharmacie pour le compte de ses parents ou de son conjoint, si ceux-ci sont en incapacité de se déplacer ? de la situation de l'aidant ? L'achat de nouveaux lecteurs de cartes Vitale biométriques pose également un problème financier et technique non négligeable. Bien sûr, le développement de la biométrie constitue une opportunité pour les pouvoirs publics en termes de sécurisation de l'identité des individus et de rationalisation de l'action administrative.

Le stockage centralisé des données biométriques collectées constituerait une base de données particulièrement exposée aux risques de cybercriminalité. Je m'étonne, par ailleurs, que l'auteur du texte n'ait pas cru bon d'insérer le nécessaire avis de la CNIL sur le traitement prévu des données.

Son appel du 15 novembre sur les enjeux de la reconnaissance faciale doit nous faire prendre un peu de hauteur. Revenons au texte lui-même. Je comprends bien qu'il faille sauver cette fausse bonne idée par le biais d'une expérimentation, mais il serait étrange de se lancer dans une telle aventure sur le fondement d'une suspicion de fraude massive, laquelle n'est même pas démontrée par les données présentées par les organismes compétents. J'ai bien peur que nous parlions un peu dans le vide, mes chers collègues. Quel est, d'ailleurs, l'avis des praticiens et des professionnels de santé, qui devraient, comme vous l'affirmez, être confrontés quotidiennement à cette problématique ? Avons-nous recueilli leur point de vue ou déclenché une enquête nationale sur cette question épineuse pour formuler une réponse législative adéquate ? Sont-ils d'accord avec le dispositif proposé et acceptent-ils d'endosser le rôle de contrôleur d'identité ?

ainsi que contre la fraude fiscale, au lieu de pointer l'élément le plus infime, qui instille une suspicion malsaine. L'emballement médiatique à la suite des annonces des auteurs du récent rapport parlementaire démontre bien l'appétence pour le sujet de certains entrepreneurs politiques, décidés à faire passer les étrangers résidents,

En premier lieu, un tel dispositif rendrait extrêmement difficile, voire impossible, la circulation de cartes frauduleuses. Comme le rappelaient les journalistes de dans un article consacré au sujet en 2016, les 100 millions de cartes pointés du doigt par l'IGAS en 2004 étaient non pas des cartes frauduleuses, mais des cartes en surnombre. Ce surplus de cartes Vitale résultait en effet d'un changement de régime ou de région qui entraînait presque systématiquement la création d'une nouvelle carte, sans restitution de la précédente. Ces anciennes cartes existent toujours, mais sont devenues inactives. Par ailleurs, les contrôles effectués dans le système d'information bloquent les flux portés par les fausses cartes.

de vue théorique, je suis tenté de répondre par l'affirmative puisque falsifier des empreintes digitales est compliqué et nécessite une certaine technicité. De plus, le système biométrique n'est pas nouveau : il existe déjà pour les cartes d'identité et les passeports. Néanmoins, c'est justement cette analogie qui suscite un certain nombre d'interrogations.

? Comment contrôler les patients qui ne peuvent se faire soigner qu'à domicile ? Au-delà des infrastructures nécessaires, il faudrait également mobiliser du personnel pour contrôler l'utilisation des appareils de lecture par les usagers, afin d'éviter que la carte ne serve à un bénéficiaire autre que son titulaire. Enfin, il faudra également renouveler intégralement l'ensemble des cartes Vitale actuellement en circulation. La proposition de loi, dans sa rédaction initiale, posait donc des problèmes importants en termes de coûts de fabrication, d'achat de matériel et de mobilisation de personnel, qu'il paraissait extrêmement difficile d'évaluer avec précision.

En somme, les membres du groupe RDSE ne sont pas opposés au texte proposé par la commission des affaires sociales et voteront majoritairement en faveur de son adoption.

Il est également indispensable de se saisir du problème de la fraude fiscale, dont le coût est estimé entre 60 et 100 milliards d'euros par an, et sur laquelle nous attendons les résultats du rapport de la Cour des comptes commandé par le Premier ministre en début d'année. La lutte contre les fraudes de toutes natures doit constituer une priorité, car elles pèsent lourdement sur les finances publiques et représentent, très probablement, un manque à gagner de plus de 100 milliards d'euros pour l'État, pour les

Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence, dans la tribune d'honneur, d'une délégation de sénateurs du Cambodge, conduite par M. Mom Chim Huy, président de la commission de la culture et président du groupe d'amitié. La délégation est accompagnée par notre collègue Catherine Procaccia, membre du groupe d'amitié France-Cambodge, qui a accueilli hier la délégation dans son département du Val-de-Marne. Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt que la délégation porte à notre institution, dans le cadre des relations anciennes et fructueuses entre nos deux assemblées et en tant que partenaires au sein de la Francophonie. Mes chers collègues, en votre nom à tous et au nom du Sénat, permettez-moi de souhaiter à nos homologues du Sénat cambodgien la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour. Nous reprenons

qui aurait pu conforter la proposition de loi déposée par notre collègue Philippe Mouiller tendant à instituer une carte Vitale biométrique, afin de lutter contre l'utilisation de vraies cartes Vitale par des personnes qui n'en sont pas titulaires.

En pratique, la carte Vitale biométrique serait délivrée après vérification de l'identité du titulaire et de la validité de sa carte d'assurance maladie ; les empreintes digitales seraient stockées sur une puce. Les professionnels de santé seraient chargés de vérifier l'identité du détenteur de cette nouvelle carte. La mise en place du dispositif s'accompagnerait d'un traitement de données spécifique, intégrant notamment l'image numérisée des empreintes digitales. Reste, mes chers collègues, que cette proposition de loi soulève plusieurs interrogations. D'abord, une expérimentation de la e-carte Vitale est en cours depuis mai dernier, et une généralisation de la version dématérialisée de la carte Vitale sur smartphone est prévue à partir de 2021. carte rejoindra ainsi la technologie de la carte européenne d'assurance maladie, déjà dématérialisée. Preuve que les systèmes biométriques commencent à être dépassés. Actuellement expérimentée par deux caisses primaires d'assurance maladie et deux caisses de mutualité sociale agricole, la e-carte Vitale a été présentée par la CNAM et le GIE Sesam-Vitale comme une bonne solution, : elle assure l'actualisation des droits en donnant la possibilité aux professionnels de santé de vérifier les droits du bénéficiaire en temps réel, un service de consultation des droits interrégimes intégré au logiciel de gestion administrative des patients elle garantit que le titulaire de la carte en est bien le détenteur, grâce à une identification biométrique réalisée préalablement, au moment de l'enrôlement. Mes chers collègues, le décret de mise en application de l'expérimentation de l'e-carte d'assurance maladie, publié au le 27 mai dernier, prévoit qu'un rapport d'évaluation sera rendu au plus tard deux mois avant le terme de l'expérimentation, c'est-à-dire en mars prochain. lors, quel serait l'intérêt de voter aujourd'hui une expérimentation de la carte biométrique ? Outre que le rapport sur l'e-carte Vitale sera rendu dans quatre mois, l'expérimentation de la carte biométrique soulèverait de nombreuses

les professionnels de santé n'adhèrent pas au projet. S'agissant, premièrement, de la protection de la vie privée et des données personnelles, le RGPD étant d'application directe et s'imposant à la loi, une disposition prévoyant l'obligation d'effectuer une analyse d'impact préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données pose un problème de conformité. En ce qui concerne la CNIL, bien que le système d'informations que supposerait le traitement des données biométriques soit motivé par une mission d'intérêt public, il soulèverait des interrogations en matière de proportionnalité de l'outil retenu, ainsi que de sécurité. Le traitement de données sensibles peut être envisagé lorsqu'il sert un objectif d'intérêt public, si et seulement si l'insuffisance manifeste des traitements existants est démontrée. Compte tenu de l'expérimentation en cours de l'e-carte Vitale et de ses effets en matière de lutte contre la fraude, l'objectif visé par la création d'une carte Vitale biométrique serait considéré comme satisfait par les traitements de données existants. proposition de loi prévoit le stockage centralisé des données biométriques collectées. Cette base de données serait particulièrement exposée aux risques de cybercriminalité. Nul besoin d'être Besson ou Spielberg pour imaginer des scénarios catastrophes surcroît, le risque est amplifié par l'exigence d'une durée de conservation de dix ans prévue dans le texte, alors que la CNIL estime la durée de conservation de trois

avec l'introduction d'une donnée biométrique, pour une masse financière de 900 millions d'euros ; enfin, le coût de l'équipement de l'ensemble des professionnels de santé est estimé à 60 millions d'euros- sans compter le développement nécessaire de logiciels adaptés par tous les éditeurs de cartes Vitale.

déposée par nos collègues Philippe Mouiller, Bruno Retailleau et Alain Milon et cosignée par l'ensemble des membres du groupe Les Républicains. Qu'est-ce que la biométrie ? La science de l'analyse des caractéristiques physiques et comportementales propres à chaque individu. individu. La biométrie permet d'identifier et d'authentifier une personne sur la base d'un ensemble de données reconnaissables, vérifiables, uniques et spécifiques. Plus précisément, l'identification biométrique consiste à déterminer l'identité d'une personne, donc de répondre à la question : qui est-elle ? Quant à

Cette proposition de loi s'inscrit par conséquent dans une logique d'authentification de l'individu. La volonté d'accroître le contrôle des identités fait suite au constat édifiant d'une explosion de la fraude à la sécurité sociale ces dernières années.

que la sienne, le tribunal de Strasbourg ayant estimé que l'administration savait qu'une incertitude entourait son identité ... Ce type de situations accentue la défiance des bons élèves à l'égard de notre système de solidarité. Pour en revenir au cas particulier de la fraude à la sécurité sociale, on estime à 261 millions d'euros les préjudices détectés et stoppés pour la seule année 2018. À titre de comparaison, ces préjudices s'élevaient à 120 millions d'euros en 2011. Face à ce constat et devant ce coût élevé, et parce que chaque euro fraudé est un euro d'argent public non perçu par l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie a renforcé la mobilisation de ses agents pour lutter contre cette tendance forte. Toutefois, les failles de notre système sont immenses. Malgré tous ces efforts, la fraude à l'assurance maladie perdurera tant que l'authentification ne sera pas sécurisée.

La mise en place d'une carte Vitale biométrique pose nécessairement certaines questions, notamment sur le plan pratique. Ainsi, les pharmaciens d'officine n'ont pas toujours les patients devant eux au moment où ils délivrent les médicaments. Ce cas particulier résume à lui seul les difficultés auxquelles pourraient être confrontés certains professionnels de santé en cas de mise en place de ce dispositif. L'expérimentation proposée par la rapporteure, Catherine Deroche, doit permettre de répondre à ces interrogations.

et rompt notre pacte social. Il convient d'agir sans délai à son encontre et de mieux protéger notre système contre les fraudeurs.

à la qualité du débat public. Au reste, j'ai récemment publié un rapport sur la fraude documentaire des personnes nées à l'étranger, c'est-à-dire la fraude aux documents utilisés pour obtenir une immatriculation à la sécurité sociale, dont le préjudice financier

Les travaux de Nathalie Goulet et Carole Grandjean ont mis en lumière que le nombre de cartes Vitale en activité excède de plusieurs millions celui des bénéficiaires couverts par les caisses de sécurité sociale. La proposition de loi dont nous débattons tend à apporter une réponse intéressante en matière de lutte contre la fraude aux prestations d'assurance maladie. Le rapport soulève plusieurs difficultés,

C'est pourquoi la rapporteure a proposé d'instaurer un délai d'expérimentation d'un an qui nous permettra de procéder à des évaluations, d'identifier les éventuelles difficultés techniques et juridiques

l'idée ne date pas d'aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, alors candidat, l'avait soutenue en 2012 ; puis, dès 2015, certains de nos collègues avaient déposé une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale,

On peut considérer qu'il y a fraude à l'assurance maladie de la part des assurés dès lors qu'il y a, chez le fraudeur, conscience de percevoir des indemnités injustement versées. Les sanctions encourues sont lourdes : le code de la sécurité sociale prévoit une amende pouvant atteindre 5 000 euros. Si la circulation de fausses cartes Vitale relève davantage du mythe, l'utilisation de cartes Vitale par des personnes qui n'en sont pas les titulaires apparaît, en revanche, comme une évidence, de même que l'utilisation de leur carte Vitale par des personnes ne résidant plus en France.

Je rappelle que, pour bénéficier des prestations sociales, il faut répondre à des conditions d'existence, de résidence et de ressources. La CNAM mène chaque année des campagnes de contrôle de la situation des assurés sur la résidence desquels elle ne dispose pas d'informations récentes ; entre entre janvier 2018 et mars 2019, elle a ainsi procédé à la fermeture des droits de 130 000 personnes. Face à un préjudice lié à la fraude qui se situerait aux environs de 120 millions d'euros, de 120 millions d'euros, nos deux collègues parlementaires ont présenté un certain nombre de propositions, notamment la limitation à deux ans de la durée de validité des cartes Vitale, avec reconduction sous conditions.

termes, on inclurait dans la puce les données biométriques du patient, comme ses empreintes digitales. Cet enregistrement serait accompagné des informations relatives à l'identité, au sexe, à la taille et à la couleur des yeux du titulaire, ainsi que de sa photographie. Ce dispositif nécessitera la mise en oeuvre d'un traitement des données à caractère personnel, et seuls les agents habilités des organismes de sécurité sociale pourront accéder à ces informations, conservées pour une durée maximale de dix ans. que la mise en place d'une telle carte biométrique pose un certain nombre de difficultés pratiques. D'abord, le recueil des empreintes risque d'être coûteux pour les organismes sociaux et l'État. Certes, le texte prévoit d'y remédier par une taxe additionnelle sur le tabac ; mais il y a fort à parier que le relevé des empreintes sera assuré pour partie par les collectivités territoriales, avec des conséquences financières Ensuite, l'expérimentation en cours de la carte Vitale dématérialisée le téléphone mobile, la e-carte, qui fait aussi intervenir des éléments biométriques, mais seulement sur la base du volontariat, doit être poursuivie, afin de mesurer l'adhésion de la population à un tel dispositif. Enfin et surtout, inscrire des données biométriques sur la carte Vitale n'aura d'intérêt que si elles sont vérifiées au moment de l'utilisation de celle-ci, pour éviter toute usurpation d'identité. Or si l'on peut imaginer des lecteurs d'empreintes digitales dans les hôpitaux, cette solution semble difficilement applicable dans les cabinets de médecins de ville, surtout en milieu rural. Les médecins pourraient refuser de jouer les contrôleurs, le contrôle des droits des usagers n'ayant pas vocation à entrer dans les missions des personnels de santé, déjà surchargés de démarches administratives.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous avons certainement tous à l'esprit des exemples d'utilisation frauduleuse de cartes Vitale racontés par des personnels soignants de notre connaissance. La fraude plus fréquente et assurément la plus visible depuis qu'une photo figure concerne les personnes soignées qui ne sont pas réellement les titulaires de la carte Vitale présentée. L'objectif de ce nouvel outil, la carte Vitale biométrique, est donc louable. Il s'agit de remédier à ces abus

m'inspire, à titre personnel, quelques inquiétudes et quelques questionnements. D'une part, la mise en oeuvre de la carte Vitale biométrique ne répondra naturellement qu'à une petite partie de la fraude actuellement constatée : la fraude ayant trait à l'identité du patient. ce type de fraude, d'après le récent rapport de Nathalie Goulet et Carole Grandjean, ne représente qu'une partie infime des fraudes à la sécurité sociale. D'autre part, la généralisation d'un tel outil biométrique représentera indubitablement un coût important. Il convient

la mise en place de cet outil ne saurait être efficace que si le contrôle de l'identité se fait réellement. Concrètement, y aura-t-il des scanners d'empreintes digitales chez les médecins, dans les hôpitaux, les pharmacies et les autres lieux d'utilisation de la carte Vitale ? l'adhésion du personnel médical est indispensable pour rendre efficace ce nouvel outil, les médecins, nous le savons, préfèrent soigner plutôt que de procéder à des vérifications d'identité.

en un ? Attentatoire au principe de solidarité qui fonde notre système de protection sociale depuis l'après-guerre, la fraude sociale doit naturellement être combattue. Par ailleurs, dans le contexte économique et social difficile que nous connaissons depuis plusieurs années, nous avons l'obligation de nous atteler à éliminer toutes les formes de fraude qui réduisent nos capacités budgétaires. que le rapport Goulet-Grandjean décrit une fraude désormais variée, généralisée, parfois organisée. À cet égard, si la prévention reste l'une des meilleures armes pour lutter contre la fraude, les fraudeurs sont de plus

en raison à la fois de son caractère frontalier, qui favorise une fraude transfrontalière forte, dont le rapport Goulet-Grandjean fait état, et du fait qu'elle accueille nombre de migrants en provenance de tous les pays d'Europe et que nous renvoient gentiment nos amis d'outre-Rhin. La discussion

Totem, car la question symbolise le manichéisme malsain de ceux qui opposent la France du travail à une prétendue France des assistés, sans considérer les chiffres du non-recours, qui infirment une telle présentation simplificatrice.

Le Gouvernement a le mérite de se pencher sur cette problématique, qui constitue une entorse à notre contrat social. Il a ainsi confié une mission à notre collègue Nathalie Goulet et à la députée Carole Grandjean, dont les travaux soulignent notamment l'existence de près de 5 millions de cartes Vitale en surnombre, de cartes Vitale en surnombre, résultat de doublons administratifs et de cartes désactivées. Si ce problème avait déjà été soulevé en 2013, l'impossibilité de chiffrer les fraudes et d'éclaircir les conditions de maintenance et les contenus des fichiers laisse aux travaux de nos collègues parlementaires un goût d'inachevé. Il est donc désormais nécessaire d'identifier les doublons, de chiffrer le montant de la fraude et de répondre à ce défi, afin de ne pas le laisser aux mains des rhinocéros au cuir épais, à la vue basse et toujours prêts à charger, pour reprendre la juste image de Claude Malhuret.

La possibilité de sécuriser l'attribution aux bénéficiaires de l'assurance maladie d'une carte Vitale biométrique constitue, à l'évidence, un moyen sérieux de lutter contre cette fraude, qui représente une part importante de la fraude aux prestations d'assurance maladie.

Toute fraude doit, par nature, être combattue, quelle qu'en soit la raison, car elle affaiblit le pacte social en détournant une partie de l'argent des cotisants de sa finalité. J'ai entendu évoquer une stigmatisation

par les caisses de sécurité sociale. Par ailleurs, un rapport de l'IGAS a clairement établi que la détention de plusieurs cartes Vitale encore valides permet sans difficulté à un nombre important de personnes de bénéficier indûment de prestations avec un autre nom.

Gouvernement ? L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale conditionne déjà la validité de la carte Vitale au droit de bénéficier de prestations au titre d'un régime d'assurance maladie et aux mises à jour concernant un changement de régime ou des conditions de prise en charge. La solution proposée conduirait à produire davantage de cartes, accroissant le coût et les difficultés de gestion tant pour les assurés que pour les professionnels de santé qui en ont besoin pour facturer les soins. Concernant

Compte tenu de l'importance de la transparence dans ce domaine technique, je ne suis pas opposée à ce qu'un rapport puisse déterminer les actions menées en la matière et, le cas échéant, proposer des améliorations, notamment pour les petits régimes qui n'ont pas toujours la puissance d'action du régime général.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Je tiens tout d'abord à remercier mon groupe d'avoir bien voulu consacrer son droit de tirage à ce beau sujet et de m'avoir confié ce rapport. Je tiens ensuite à remercier la présidente de la mission, Michèle Vullien, de notre relation de travail riche, franche et constructive. également à remercier chacun des membres de cette mission de leur implication dans nos travaux. Enfin, je tiens à remercier l'équipe d'administrateurs qui n'a pas ménagé ses efforts pour aboutir au riche rapport dont nous débattons aujourd'hui. La gratuité des transports : fausse bonne idée ou révolution écologique et sociale des mobilités Telle est la problématique que nous avons posée pour étudier ce sujet popularisé, entre autres, par le choix opéré par la métropole de Dunkerque, et de plus en plus présent dans le débat public à mesure que les élections municipales approchent. Après plus de quarante-sept heures d'auditions, les réponses de nombreuses collectivités, une consultation en ligne qui a récolté 10 500 contributions-un record et une preuve, si besoin en était, de l'intérêt du sujet pour nos concitoyens-, notre rapport se veut un outil d'aide à la décision. La gratuité d'un service public pour ses usagers est un sujet d'ordre quasi philosophique, dont chacun peut s'emparer aisément, et qui enflamme facilement les débats ou les discussions. On ne se pose plus la question de la gratuité de l'école publique ou celle de l'accès aux soins essentiels.

La question est donc la suivante : notre République doit-elle assurer un droit universel à la mobilité, comme elle assure un droit universel à l'éducation ou à la santé ? C'est un vaste débat qui agite les passions et qui voit trop souvent s'affronter des positions de principe, pas toujours étayées, pas toujours éclairées. Que l'on soit pour ou contre le principe de la gratuité, on assiste souvent à un florilège d'idées reçues et de lieux communs que le premier objectif de ce rapport était d'éprouver. Je ne citerai que deux exemples. Non, la gratuité des transports ne conduit pas aux incivilités ou à une dégradation des équipements. Et non, la suppression de la billettique et des contrôles ne suffit pas à compenser les pertes de recettes. de l'une de nos premières recommandations : dépasser les positions de principe et les idées reçues pour débattre des faits, des chiffres et des réalités de chaque territoire et de chaque réseau. Le rapport dresse donc un état des lieux de la mise en oeuvre de la gratuité des transports en France- cela concerne vingt-neuf communes à ce jour -et dans le monde. Il trace des perspectives pour repenser la mobilité collective au XXIsiècle. Le premier constat est sans appel : nous n'avons que très peu de recul sur le sujet. Les expériences françaises et internationales sont assez rares et les études scientifiques le sont encore davantage, notamment pour déterminer clairement le type de report modal qu'implique la gratuité. Les données que nous avons collectées sont parcellaires et ne permettent pas de tirer des conclusions irréfutables. C'est pourtant une nécessité de pouvoir se fonder sur des études précises pour évaluer objectivement le bilan environnemental de la gratuité. ce rapport, nous proposons de mettre en place un observatoire de la tarification des transports pour accumuler des données statistiques et scientifiques à même d'éclairer la décision publique. Cela étant, l'étude de l'Agence de et l'étude plus récente réalisée par la ville de Dunkerque semblent montrer assez nettement que la gratuité des transports est une mesure sociale très efficace. Là où elle a été mise en place, la fréquentation des bus a grimpé : on observe une hausse du nombre des usagers de 23 % à Niort en deux ans et de près de 80 % à Dunkerque en moins d'un an.

Le principal inconvénient de la gratuité est paradoxalement son efficacité. Elle oblige à se poser la question de l'offre de transport. Ainsi, dans les réseaux déjà extrêmement fréquentés- on pense naturellement à la région capitale, mais c'est le cas pour d'autres réseaux une mise en oeuvre de ce principe risquerait d'entraîner une saturation totale du réseau et, donc, une baisse de la qualité du service. Dans les grandes agglomérations qui possèdent des réseaux denses, il est nécessaire d'établir des priorités. Les questions de l'offre de transport et de sa soutenabilité dans le temps doivent prévaloir sur celle de la gratuité. C'est d'autant plus important que les réseaux ferrés des grandes métropoles sont beaucoup plus coûteux à développer et à entretenir que les seuls réseaux de bus. Cette problématique nous invite aussi à considérer que la gratuité n'est pas une fin en soi ni un but absolu. d'un outil de politique publique parmi d'autres, qui doit s'inscrire dans un projet de mobilité, un projet urbain plus vaste. Ainsi, pour toutes les villes moyennes où les réseaux sont neufs et sous-utilisés et dont les centres-villes sont de moins en moins fréquentés, la gratuité des transports, associée à une politique de revitalisation des centres-villes, est un outil extrêmement efficace, comme le prouvent les exemples de Châteauroux, de Dunkerque ou de Niort. C'est une autre recommandation du rapport que de penser la gratuité comme un levier au service d'une politique globale, et non comme un objectif à part entière. En effet, la gratuité pose fondamentalement la question du financement des transports

Alors que mon propos touche à sa fin, et avant de vous présenter les deux dernières recommandations du rapport, permettez-moi d'ajouter un commentaire plus personnel. Ma conviction est que la gratuité des transports relève d'abord d'un choix politique, plus ou moins ambitieux en fonction des territoires et des réalités locales. Pour ne donner qu'un seul chiffre, le coût consacré à l'entretien et au fonctionnement de tous les réseaux de transport en commun du pays s'élève à environ 16 milliards d'euros, somme financée par les usagers, les contribuables locaux et les entreprises.

C'est paradoxal quand on songe aux urgences sociales et écologiques auxquelles nous devons faire face. À titre personnel, je pense qu'il s'agit d'un horizon vers lequel toutes les collectivités peuvent et doivent tendre selon un rythme adapté à leurs particularités, la gratuité partielle constituant un premier pas Enfin, nos travaux nous conduisent à deux réflexions plus larges : l'une sur la mobilité entre zone rurale et zone urbaine, l'autre sur la « démobilité ». Attention aux distorsions entre des territoires peu ou pas dotés en transports en commun et des centres urbains disposant de l'ensemble des services, qui sont de surcroît gratuits. se pose est celle de notre projet urbain, de la taille de nos villes, de l'étalement urbain, de la dissociation entre les zones d'activités économiques et les zones d'habitat. Alors que les centres-villes de nos communes moyennes sont en déshérence, que la transition agricole nécessite une multiplication des emplois et, donc, une forme d'exode urbain, nous sommes amenés à considérer

sénatoriale, complet et équilibré, souligne combien il importe de faire évoluer notre modèle de transport vers des mobilités plus propres et plus solidaires. Ce sont des objectifs que nous partageons tous, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour y parvenir. je précise que je préfère parler de « choix de tarification » plutôt que de « gratuité », car, comme nous le savons tous, la gratuité des services publics n'existe pas : ces services ont un coût, la question posée étant celle de la répartition de ce coût entre le contribuable et l'usager.

Une fois le débat posé en ces termes, il est particulièrement important que le Gouvernement puisse y prendre part, et ce au moment même où le projet de loi d'orientation des mobilités est sur le point d'aboutir. Votre travail met parfaitement en évidence les trois objectifs, parfois difficilement conciliables, auxquels doit répondre une politique tarifaire : garantir le droit au transport pour tous, favoriser une politique de report modal et, enfin, couvrir une partie des coûts de production du service. La tarification relève de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, à ce titre, d'un choix politique fait en responsabilité par les élus locaux. Ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins de leurs concitoyens, si bien que l'État n'a pas à décider à leur place.

Pour autant, vous le savez, d'autres solutions existent pour atteindre cet objectif. La tarification solidaire en fonction des revenus ou du statut, mise en place par de nombreuses autorités organisatrices, apparaît, en termes de pouvoir d'achat, comme une alternative efficace pour répondre à la problématique de mobilité des populations les moins aisées. aisées. Elle me semble également plus égalitaire, car elle est fondée sur la capacité financière des usagers. C'est d'ailleurs le choix que fait la grande majorité des collectivités locales, qui aident les usagers des transports publics sous condition de ressources, les étudiants, aux côtés des entreprises qui contribuent au financement de l'abonnement de leurs salariés. De plus, la question de la tarification ne doit pas monopoliser le débat et masquer les autres enjeux en matière de solidarité et d'accès à la mobilité. Pour les publics les plus fragiles, un accompagnement à la mobilité et des solutions spécifiques sont nécessaires.

Par ailleurs, comme la consultation que vous avez conduite l'a bien montré, l'enjeu en termes d'accès à la mobilité réside d'abord et avant tout dans le développement d'une offre utile. Le premier frein à la mobilité sur un territoire, c'est l'absence d'offre adéquate. La question de la tarification ne vient qu'après.

Concernant l'enjeu écologique, le manque d'évaluations à notre disposition doit nous conduire à rester prudents sur l'incidence de la gratuité pour l'usager en matière de report modal de la voiture particulière vers les transports en commun. On peut toutefois relever que les reports modaux observés dans les territoires sont en général le fruit d'une politique globale de mobilité qui dépasse le seul enjeu de la tarification. Celle-ci combine une politique visant à améliorer l'offre de transport et une politique vous noterez la plus grande sensibilité des associations d'usagers aux notions de desserte ou de ponctualité qu'à celle de gratuité. Par ailleurs, il convient de déployer une politique de régulation de l'usage de la voiture, notamment au travers du stationnement. En revanche, la gratuité pour l'usager permet indiscutablement d'améliorer la fréquentation des services de transport existants, en fidélisant certains usagers et en attirant d'autres publics qui ne sont pas captifs du confort ou de la rapidité de la voiture.

Enfin, si l'incidence de la gratuité pour l'usager en matière sociale et écologique prête à débat, il n'en est pas de même sur le plan économique, puisque la perte de ressources pour la puissance publique est, pour le coup, tout à fait tangible.

la gratuité est mise en oeuvre, elle est financée par le contribuable local : les employeurs au travers du versement transport, qui deviendra bientôt le versement mobilité, et les habitants au travers de la fiscalité locale. Si certains territoires peuvent s'appuyer sur un réel dynamisme économique avec la présence de grandes entreprises pour financer la part de l'usager, ce n'est pas le cas de tous. Ce n'est donc pas un hasard si les réseaux gratuits pour l'usager, une trentaine aujourd'hui en France, sont pour la plupart de taille modeste, avec un taux de fréquentation souvent plus faible que la moyenne.

les exemples étrangers sont une source d'enseignement, puisque certaines villes ont rétabli une tarification pour faire face aux besoins de financement liés au développement de l'offre. En conclusion, mesdames, messieurs les sénateurs, vous aurez compris au travers de mon intervention que le Gouvernement, tout en respectant le choix souverain des collectivités locales, souhaite d'abord développer les offres de mobilité partout dans notre pays et pour tous nos concitoyens. Le premier facteur d'exclusion ou de discrimination, c'est non pas la tarification, mais l'offre. Ainsi, c'est d'abord en démultipliant les offres concrètes de mobilité que nous répondrons à la principale demande de nos concitoyens. Vos travaux vont nous permettre d'échanger sur ces sujets au cours de débats qui s'annoncent, j'en suis certaine, riches et constructifs. chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

sensibilité politique, mais pas seulement. Nous estimons aujourd'hui et plus que jamais, alors que l'impératif climatique devient incontournable, que la gratuité, en complément

ce qui correspond à près de 16 milliards d'euros chaque année, soit davantage que les 12,6 milliards d'euros que représentaient les dépenses pour l'entretien et le fonctionnement des transports publics urbains en 2018.

Plutôt que d'essayer de répondre à la dictature du court terme, en oubliant l'intérêt général, rappelons-nous que ce type de dispositif est une réponse de long terme et qu'il doit s'intégrer dans une politique globale des transports collectifs et de la mobilité. nous le démontre le rapport, la gratuité totale n'est applicable que dans des collectivités de taille réduite, ayant un réseau unique et sous-utilisé. Pour les autres, notamment les métropoles, l'adaptabilité peut être envisagée grâce à certaines mesures de gratuité partielle, telles que

La mise en place de toutes ces solutions modulables en fonction du territoire nécessite des recettes : il s'agit de la question centrale, car celles-ci diffèrent en fonction du type de collectivité et de la localisation. Au moment où des solutions plus écologiques en matière de transport sont étudiées, où certains développent de nouveaux projets de mobilité soutenables pour les collectivités, il nous faut mieux outiller les acteurs de la mobilité, afin de répondre aux attentes des citoyens et aux besoins de tous les territoires. Chaque offre de mobilité est spécifique, apporte sa richesse et sa singularité. Chacun de nos territoires est concerné, qu'il soit urbain, périurbain ou rural. Madame la secrétaire d'État, afin que ce dispositif ne devienne pas une fausse bonne idée et qu'il puisse s'appliquer quel que soit le territoire- je pense surtout aux zones rurales -, pourriez-vous nous détailler les outils que le Gouvernement envisage de proposer aux autorités organisatrices de la mobilité ?

Les autorités organisatrices de la mobilité restent libres de leur politique tarifaire, de l'appréciation de leurs marges de manoeuvre financières et fiscales. Vous l'avez également mentionné, c'est bien une politique de long terme que ces autorités doivent conduire.

Mais il est des territoires où cette question passe après celle de la réalité et de la qualité des transports, tant ceux-ci sont déficients. Je pense en particulier aux difficultés que rencontrent les travailleurs transfrontaliers du nord de la Lorraine, qui se rendent chaque jour dans le Grand-Duché de Luxembourg. Ils se heurtent à d'énormes problèmes de circulation, car tous les réseaux sont saturés, y compris ceux des transports collectifs.

de l'impôt sur le revenu des travailleurs frontaliers et que, pour l'heure, ils n'envisagent aucune rétrocession fiscale, à la différence de ce qui prévaut avec la Belgique, par exemple

En matière de voyageurs, il faut bien reconnaître qu'il est très difficile d'intéresser les autorités du Luxembourg au sort des travailleurs frontaliers français, comme le démontre la situation des TER français qui ne pourront plus franchir la frontière à Thionville à partir du 1janvier prochain. L'État continue à se mobiliser, et les secrétaires d'État Jean-Baptiste Djebbari et Amélie de Montchalin ont encore écrit tout récemment au ministre luxembourgeois chargé Les participations luxembourgeoises sont d'ailleurs rarement désintéressées. Ainsi, les investissements dans les TER, soutenus par le Luxembourg à hauteur de 120 millions d'euros en application d'un protocole intergouvernemental de mars 2018,

Enfin, en matière de développement économique, vous l'avez rappelé, le principe d'une compensation financière des États où travaillent les frontaliers au profit des États où ceux-ci résident a été validé par le Conseil de l'Europe le 29 octobre dernier.

La liste est longue des services proposés à la population qui font l'objet de débats apparaissant ou réapparaissant à la veille des élections municipales : gratuité de l'eau, gratuité de la restauration scolaire, gratuité de la piscine, gratuité des transports, et j'en passe.

L'incidence, ou plutôt le bénéfice environnemental de la gratuité n'est pas avéré. Elle ne favorise qu'un report modal très limité : le nombre de voitures ne diminue pas ou très peu, le transfert s'opérant du vélo et de la marche à pied vers les transports en commun. L'impact financier est préjudiciable à l'autorité organisatrice et, de fait, aux entreprises qui paient le versement mobilité.

Comme le montre la mission d'information, ainsi que l'étude menée par le GART, l'incidence de la gratuité sur le report modal de la voiture particulière vers les transports publics reste difficile à mesurer. Les effets en termes de report modal sont généralement la conséquence d'une politique d'ensemble, visant, d'une part, à améliorer l'offre et la qualité des transports, d'autre part, à réguler l'espace, notamment à travers la politique de gestion de l'espace public ou de stationnement. Pour mieux mesurer l'impact propre de la gratuité, des outils méthodologiques adaptés pourraient être mis en place par les réseaux. Ils permettraient de mieux appréhender et objectiver le report modal. Selon certains, il semble que la gratuité ait eu peu d'effet sur ce dernier, mais qu'elle diminuerait en revanche la part du vélo et de la marche, ce qui pose évidemment question. Par ailleurs, l'aide à la décision des collectivités locales en matière tarifaire doit les amener à s'interroger sur l'équilibre entre dépenses et ressources, afin de disposer des moyens nécessaires pour répondre aux besoins. L'État soutient donc la proposition de la mission de mettre en place un observatoire de la tarification des transports pour recenser des éléments plus objectifs, notamment sur le report modal, et constituer ainsi une aide à la décision pour les choix tarifaires des élus locaux.

comment accompagner les territoires les plus fragiles, dès lors que, dans le projet de loi Mobilités, vous avez refusé les dispositifs proposés unanimement

Les communautés de communes qui prendraient volontairement la compétence disposeraient ainsi d'une recette dynamique, permettant d'asseoir le développement de services de mobilité alternatifs à des services collectifs réguliers. Par ailleurs, l'État, au travers de la démarche France Mobilités, accompagne les territoires qui le souhaitent. Cet accompagnement passe par des appels à projets, comme vous le savez, avec des financements dédiés pour la prise de compétence, notamment au travers de cellules régionales d'appui à l'ingénierie. Mais le projet de loi d'orientation des mobilités, c'est également un engagement de l'État d'investir 13,4 milliards d'euros dans les infrastructures de transport sur l'ensemble du quinquennat, partout sur le territoire. Cet effort, significatif, est sans précédent ; il est évidemment nécessaire.

dans cet hémicycle, j'alerte sur le cauchemar que vivent les usagers du RER francilien et je rappelle que notre système de transport est à bout de souffle, au bord de l'explosion. Chaque fois, on m'explique que le Gouvernement investit bien plus qu'avant, progresse sur le projet du Grand Paris, finance les transports du quotidien. C'est sans doute vrai, mais ces mesures sont clairement insuffisantes pour répondre à la lourde crise à laquelle nous sommes confrontés et que tous les gouvernements ont systématiquement minimisée.

Mais où sont les trains RER et les bus qui permettront à des centaines de milliers d'habitants de la grande couronne de laisser leur voiture pour prendre les transports en commun ? Le Grand Paris Express, même s'il était achevé dans je suis optimiste -, n'arrive pas jusqu'aux départements de grande banlieue et ne complétera donc pas l'offre du RER. Aucune mesure à la hauteur de ce défi gigantesque n'est prévue. Réveillons-nous ! Nous ne parvenons déjà pas à gérer la situation actuelle. Ces dernières semaines, encore, l'accélération des dysfonctionnements au moment des heures de pointe a bloqué des centaines de milliers de personnes sur les quais de nos gares. Les trains sont supprimés ; ils sont sans cesse en retard ; ils sont tellement bondés qu'il faut parfois en laisser passer deux ou trois pour pouvoir monter dans une rame. Les usagers ne demandent pas en priorité la gratuité des transports. Ils savent bien que les services ont un coût et qu'ils les paieront toujours d'une manière ou d'une autre. Ce qu'ils demandent, c'est tout simplement des transports qui fonctionnent ! Ils exigent de ne pas être entassés dans des wagons bondés. Ils veulent juste arriver à l'heure le matin au travail ou le soir pour récupérer leurs enfants à la crèche. leurs enfants à la crèche. C'est maintenant qu'il faut agir et créer des transports légers pour couvrir les besoins, très importants, des 4,5 millions d'habitants de la grande couronne parisienne. Qu'ils soient payants ou gratuits, s'ils fonctionnent, nous les prendrons ! La parole est à Mme la secrétaire

nombreuses études de cas confirment les prédictions de la théorie en économie des transports. Les villes ayant expérimenté une telle mesure n'ont pas observé de réduction significative de la pression automobile ni de leurs externalités. Le report modal a été systématiquement inférieur aux attentes des décideurs publics. En général, cette mesure a été associée à une augmentation de l'utilisation des transports publics provenant principalement d'un report modal depuis des modes actifs, comme la marche ou le vélo, de nouveaux trajets qui n'étaient pas effectués auparavant et d'une hausse de l'attractivité territoriale des villes concernées. Nous Nous savons que la réduction de la pression automobile passe nécessairement par un changement de paradigme, qui induit une modification du coût relatif des modes de transport. Un tel changement implique de penser conjointement la tarification des transports en commun et de l'automobile.

Différentes contributions suggèrent que les modalités de mise en oeuvre de cette tarification, comme le péage cordon, le péage de zone ou le péage sur le stationnement, jouent un rôle important en termes de performances. À titre d'exemple, des simulations réalisées pour Paris suggèrent des gains importants de bien-être, dont l'ampleur dépend de la technologie choisie. Enfin, il convient de rappeler que la tarification ne constitue pas le seul outil en mesure de modifier le coût relatif des différents modes de transport. La réduction de la pression automobile devrait être envisagée dans une approche globale de la mobilité urbaine, incluant, outre la réflexion sur la tarification des différents modes de transport, la question de l'espace laissé à l'automobile- nombre de bandes de circulation, zones accessibles, etc. -, de l'espace laissé aux autres modes de transport- transports en commun, mais aussi marche ou vélo -et la promotion d'un usage plus efficace de la voiture à travers la promotion du covoiturage et de l'auto partagée.

Les territoires sur lesquels on observe du report modal de la voiture individuelle vers d'autres modes de transport sont ceux qui ont développé, à la fois, une offre de services de mobilité diversifiée et de qualité, et une politique de régulation de la voiture, notamment par le biais du stationnement payant. La mise en oeuvre au 1 janvier 2018 de la dépénalisation du stationnement souhaitée par de nombreuses collectivités permet aujourd'hui d'utiliser ce levier pour travailler sur la place de la voiture individuelle dans les villes. Par ailleurs, plusieurs grandes collectivités se sont engagées dans la mise en place de zones à faible émission,

Cela nous montre simplement qu'il faut trouver un juste équilibre entre les contraintes et les mesures d'incitation positive. Ainsi, la mission suggère de réfléchir à d'autres solutions de mobilité, notamment les mobilités partagées, qui sont très encouragées au travers du projet de loi Mobilités. à se saisir du principe de la mobilité vue comme un service, une approche intégrée permettant à l'usager de disposer d'une information, d'une billetterie, voire d'une tarification qui combine tous les modes, indépendamment du territoire et de l'organisateur du service. Les autorités organisatrices de transports pourront ainsi développer des tarifications à l'usage, mixant toutes les formes de mobilité disponibles avec une facture en fin de mois, y compris les vélos ou les voitures partagées en libre-service. Par ces actions, le Gouvernement entend ouvrir le champ des possibles pour améliorer les solutions de mobilité sur les territoires, afin que la nécessaire transition écologique en matière de mobilité ne soit pas vécue de façon punitive par nos concitoyens. La parole est à M. Loïc Hervé. Tout en saluant le

Madame la secrétaire d'État, je vis dans un territoire, la vallée de l'Arve, qui a connu ces difficultés et qui, en même temps, doit faire face au défi de la pollution de l'air. Comment envisagez-vous d'aider les collectivités, de leur apporter des solutions

afin de répondre aux demandes légitimes des 25 % de citoyens, des 75 % de territoires dépourvus de réseau géré par une autorité organisatrice de transports, donc de solutions de mobilité organisées, la future LOM encourage les communautés de communes, qui représentent environ 20 millions d'habitants à l'échelle nationale, à exercer la compétence d'organisation de la mobilité. la mobilité. Le versement transport est sanctuarisé et devient le versement mobilité pour les collectivités qui mettront en place des services de transport collectif réguliers, afin de préserver l'acceptabilité de cet impôt assis sur la masse salariale par les acteurs économiques- vous l'avez rappelé, c'est un sujet délicat.

le versement transport est un impôt complexe pour les entreprises, cette solution conduisait à doubler le nombre d'entreprises soumises à cette imposition, ce qui les contraignait à assumer de nouvelles obligations déclaratives pour des montants très faibles. C'est pourquoi le Gouvernement n'a pas souhaité retenir cette solution et a préféré recourir à la réforme de la fiscalité locale, en substituant, comme vous le savez, de la TVA dynamique à de la taxe d'habitation moins dynamique, afin que les collectivités confrontées à un problème d'acceptabilité ou de rendement du versement transport puissent, malgré tout, disposer de ressources pour organiser des solutions de mobilité sur leur territoire. La parole est à M. Loïc Hervé, pour la réplique.

s'est appuyé sur les conclusions d'un colloque organisé en juin dernier à Nice, intitulé « Gratuité des transports publics : entre idéal et réalité compléter le rapport de la mission d'information. Le constat est assez unanime : supprimer purement et simplement le paiement des transports par les usagers est une mesure relevant du leurre, voire de la démagogie dans les territoires tendus. En effet, un service gratuit est forcément payé par quelqu'un, et la priorité pour l'usager, c'est avant tout la qualité de service. Il ne faut donc pas sacrifier la qualité à la gratuité De plus, la gratuité totale ne serait pas nécessairement au bénéfice des plus modestes, qui, bien souvent, on l'a dit, bénéficient déjà d'offres gratuites, tout comme les jeunes ou les seniors disposent de tarifs préférentiels. À cela s'ajouterait un effet d'aubaine pour les vacanciers et les touristes dans les territoires à forte attractivité touristique, comme le mien, où le réseau serait alors financé par les seuls contribuables locaux. L'offre payante est donc un levier de financement

parfois proches de la gratuité. Dans la métropole Nice Côte d'Azur, l'instauration du ticket à un euro a permis d'introduire équité et solidarité territoriale, ce ticket s'appliquant à l'ensemble des 49 communes de la métropole,

à l'heure plusieurs options : la tarification solidaire, qui permet de différencier les tarifs en fonction du revenu ou des statuts et qui apparaît comme une alternative pour répondre à la problématique de mobilité des populations les plus fragiles ; un accompagnement à la mobilité, avec la compétence mobilité solidaire et l'appui des départements et des régions par bassin de mobilité ; le développement d'une offre de qualité, considéré par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports

moins directs, inconfortables ». Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient de publier un avis sur le rapport entre travail, emploi et mobilités,

La périurbanisation a tendance à s'accentuer avec le renchérissement généralisé du coût du logement en accession à la propriété ou pour le parc locatif et social. En effet, les écarts du coût du foncier, entre le centre des grands pôles urbains et leur périphérie, incitent les actifs et actives à rechercher des logements moins chers et plus grands plus loin des zones des zones d'activité. » Les politiques d'urbanisme des années 1960 ont montré leurs limites. La pression foncière dans les centres des métropoles, concentrant des activités tertiaires, rend l'immobilier résidentiel inaccessible. lors, madame la secrétaire d'État, y a-t-il une volonté gouvernementale de mettre en place des outils de régulation, notamment la taxation des plus-values immobilières, pour financer, certes la diversification sociale du logement, mais aussi les besoins liés aux infrastructures et, de manière générale, les besoins en mobilité ?

Vous m'interrogez sur l'articulation des politiques d'aménagement et des politiques de mobilité, l'amélioration des infrastructures de transport et des services encourageant l'étalement urbain, lequel nous invite à conduire des réflexions pour diminuer ces besoins en mobilité. La mission dont nous discutons les conclusions aujourd'hui propose de poursuivre et d'élargir la réflexion sur les modes de financement de la mobilité, notamment en matière de captation des plus-values foncières. Du point de vue du Gouvernement, un travail pourrait être engagé en ce sens. Je rappelle que plusieurs mesures prévoyant l'instauration d'une taxation des plus-values immobilières liées aux infrastructures de transport ont été adoptées par le Parlement au cours des dernières années. Aucune n'a été mise en oeuvre. l'Île-de-France, la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris avait ainsi prévu l'instauration d'une taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant des projets d'infrastructures du réseau de transports du Grand Paris, mais cette disposition a finalement été abrogée par la quatrième loi de finances rectificative pour 2010. Une taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre

la part des recettes tarifaires dans les ressources des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) est significativement inférieure à celle des réseaux de transports collectifs étrangers. étrangers. En effet, en France, les employeurs sont les premiers financeurs des transports publics. À l'exception culturelle française bien connue, la France ajoute discrètement l'exception du financement des transports publics. L'apport financier des entreprises passe par deux canaux principaux : premièrement, la participation des employeurs aux frais de transport de leurs salariés, entre le domicile et le lieu de travail, pour un coût annuel de l'ordre de 900 millions d'euros pour les entreprises ; deuxièmement, le versement transport, prochainement dénommé « versement mobilité », qui est un impôt. Instauré en 1971 pour la seule région parisienne, ce versement a été progressivement étendu, de sorte que plus de 250 autorités organisatrices de la mobilité lèvent actuellement cet impôt sur les entreprises comptant plus de dix salariés. Nous constatons, au cours des quinze dernières années, une baisse généralisée de la part des usagers dans le financement des transports publics et une hausse importante du versement transport. Celui-ci représente en moyenne 47 % des ressources des AOM. Dès 2017, 67 % des AOM de plus de 300 000 habitants ont atteint le plafond. Le nombre de municipalités ou de conseils d'agglomération qui offrent le transport gratuit n'a jamais été aussi élevé. Selon le groupement des autorités responsables des transports, elles sont 29. Sous le couvert de la transition énergétique, une vingtaine de programmes électoraux proposent la gratuité totale, et plusieurs équipes sortantes y pensent à plus ou moins haute voix. Ma question, madame la secrétaire d'État, est donc la suivante : ne pensez-vous pas que l'extension de la gratuité totale risque d'amener les employeurs à contester la légitimité même d'un impôt de plus en plus éloigné de sa raison d'être initiale ? Un vieux dicton nous apprend que la cruche finit par se casser à force d'aller à l'eau ; or le versement mobilité restera indispensable pour cofinancer les investissements nécessaires à la modernisation et à l'expansion continue des transports publics. La parole est à Mme la secrétaire est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Danesi, le versement transport, effectivement, est aujourd'hui une ressource importante du financement des transports collectifs. Comme je l'ai dit plus tôt, il représente environ 44 % du coût total. C'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas l'augmenter, mais simplement le stabiliser. le stabiliser. Qu'on le veuille ou non, une gratuité entraînerait forcément un transfert de charges vers les contribuables, alors que les autorités organisatrices ont à mener des politiques de renouvellement et d'extension du réseau. Ces politiques ont un coût.

appelle donc des investissements et des dépenses de fonctionnement supplémentaires, les moyens de production, matériels et humains étant en effet dimensionnés pour absorber les heures de pointe. Ainsi, pour les plus grands réseaux, la gratuité pourrait doublement renchérir le recours à l'impôt, notamment au versement transport : par un effet prix, entraînant une baisse de ressources, d'une part, et par un effet volume, entraînant une hausse des moyens de production nécessaires, d'autre part. Comme vous le soulignez, pour la très grande majorité des réseaux de transports publics en zone dense, les besoins de mobilité sont tels que la gratuité apparaît plutôt pénalisante ; elle risquerait de remettre en cause l'équilibre subtil qui a été trouvé entre les financements de l'usager et du contribuable et de mettre en péril toute l'accessibilité du versement transport.

une vertu, celle de sortir ce débat d'une approche un peu binaire. Nous avons montré que la gratuité des transports collectifs n'est pas une idée bonne ou mauvaise en soi : tout dépend dans quel but elle est mise en oeuvre. Elle doit s'inscrire dans une stratégie locale de développement qui prend en compte les particularités du territoire et de ses habitants. Pour ma part, je préfère la notion d'accès libre aux transports. Elle illustre mieux le fait que l'accès aux transports a un coût et qu'ouvrir cet accès d'un choix de la collectivité. Cette expression permet de mieux réfléchir à des outils alternatifs : la tarification solidaire, plus ambitieuse, implique non pas la gratuité totale, mais donne la gratuité à ceux qui en ont besoin. Toutes ces mesures participent néanmoins d'une révolution sociale des mobilités, une révolution dont les effets positifs se feront sentir, à terme, pour l'ensemble des habitants : réduction de la pollution amélioration de la fluidité du trafic, etc. Ces retombées positives vont bénéficier à tous : non seulement aux collectivités et aux AOM, mais aussi à l'État, via une baisse des dépenses de santé. Pour renforcer ces externalités positives, notre rapport a mis en évidence l'éventualité de ressources alternatives à la fiscalité locale : une

Je me réfère donc à la première recommandation du rapport : « Dépassionner le débat qui souffre trop souvent de positions de principe et d'idées préconçues. » Pour revenir au fond, la décision de mettre en place la gratuité relève bien du libre choix des collectivités territoriales- et donc des autorités organisatrices de la mobilité. Des alternatives existent pour sortir de ce débat binaire. Premièrement, la tarification solidaire,

avec la compétence mobilité solidaire des AOM, soutenues par la région et le département. Troisièmement, nous devons continuer à travailler sur le développement d'une offre de mobilité. En ce qui concerne la TICPE, celle-ci est plutôt orientée vers les investissements. Elle ne me paraît donc pas une solution à ce stade.

l'évolution du climat préconisait d'atteindre une réduction de plus de 40 % des consommations d'énergie dans les transports, tout d'abord en réduisant notre usage de la voiture. Il ne s'agit pas de simples ajustements, de prendre moins souvent sa voiture. Il s'agit de changer radicalement nos modes de vie en ville. L'État et les collectivités territoriales ont une responsabilité dans le domaine des transports et de la mobilité. Les politiques doivent ainsi proposer à nos concitoyens les moyens de changer leur mode de vie, afin que la voiture ne soit pas le mode de transport prépondérant. Peu d'expériences sur la gratuité des transports collectifs sont menées à l'échelle nationale. Cependant, l'une d'entre elles retient toute mon attention, celle de l'agglomération de Dunkerque, qui compte plus de 200 000 habitants. Après avoir été expérimentée le week-end pendant trois ans, la gratuité a fini par s'étendre à la semaine. Les premières conclusions sur l'expérience dunkerquoise semblent particulièrement positives. Dans le débat des élections municipales, les maires de la métropole lilloise ont fait savoir qu'ils étaient favorables à la mise en place d'une gratuite partielle, tournée vers certains publics, notamment les jeunes, et même les très jeunes- ce à quoi je suis très favorable -, et lors des pics de pollution. La gratuité totale n'est pas possible partout. Cependant, afin de lutter contre le changement climatique, l'État et les collectivités territoriales devront mettre en place des politiques plus incitatives. Madame la secrétaire d'État, quels moyens le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre

parle essentiellement des transports en commun à l'échelle des aires urbaines. L'avant-propos précise en effet que la question des personnes vivant en zones périurbaines ou en milieu rural est une problématique plus vaste ; elle mérite un traitement à part entière, car aborder ce sujet par le prisme de la gratuité serait trop réducteur. Néanmoins, les zones périurbaines et rurales qui entourent nos agglomérations et métropoles sont parfois couvertes par des réseaux de transport émanant de la ville-centre. Le service rendu est alors fortement déséquilibré.

Les arbitrages budgétaires réalisés pour permettre cette gratuité empêcheraient, par exemple, le développement d'une meilleure offre par un réseau élargi ou un cadencement plus soutenu. En revanche, j'adhère à l'idée de la gratuité partielle. Les jeunes sont une cible privilégiée à bien des égards. Je crois à la portée éducative que pourrait revêtir ce genre de pratique, en les incitant, dès le plus jeune âge, à se déplacer différemment de leurs aînés et à adopter d'autres réflexes, plus vertueux d'un point de vue écologique. Ensuite, si le choix d'une gratuité partielle en direction des jeunes me semble pertinent, c'est aussi parce que la mobilité leur est purement et simplement imposée pendant leur scolarité ! Concernant l'exemple de Besançon et de ses communes périphériques, Grand Besançon Métropole est l'autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire. La région Bourgogne-Franche-Comté, pour sa part, organise les transports scolaires, à l'exception des zones couvertes par un réseau urbain et périurbain. La conséquence est la gratuité totale du transport scolaire pour tous les élèves du ressort de la région, la classe de terminale. En revanche, les élèves de la communauté urbaine doivent s'acquitter d'un abonnement mensuel important. Le déséquilibre, une fois encore, se fait sentir. L'absence d'une mesure nationale sur ce sujet pose le problème de l'harmonisation, qui n'est pas automatique. Je ne sais s'il s'agit d'une bonne solution ; mais, si la gratuité peut être une solution pour un cas donné ou un territoire en particulier, elle ne le sera pas forcément pour un autre. Madame la secrétaire d'État, comment le Gouvernement peut-il favoriser,

et être solidaire au sein même d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, d'une métropole, entre l'hypercentre et toutes les communes périphériques. La première solidarité consiste en une capacité à couvrir tout le territoire français et à exercer cette solidarité à l'échelle de l'agglomération. La question que vous posez est une question d'équilibre entre l'action de la région et celle des intercommunalités.

Aujourd'hui, chaque autorité organisatrice de la mobilité a mis en place une politique tarifaire plus ou moins avantageuse pour les usagers. Je ne suis pas opposé par principe à la gratuité des transports urbains ; elle peut contribuer à réduire la pollution urbaine et à donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Pour que la gratuité ait un sens, il faut qu'elle permette un réel report modal, afin d'augmenter le nombre d'usagers délaissant leur voiture au profit des transports en commun. Les études le prouvent, plus les infrastructures de transports en commun en site propre sont nombreuses, plus les usagers les fréquentent. Les usagers ne s'y trompent pas ils préfèrent à la gratuité une offre de transports collectifs payante, mais plus développée. Des questions se posent sur les conséquences de la gratuité, notamment sur la prise en compte de la hausse de la fréquentation des lignes existantes. L'équation est simple : plus de fréquentation implique un plus grand nombre de rames, plus de lignes pour atteindre l'objectif de réduction de la place de la voiture dans nos villes. Avec les modifications des modes de vie, nous pouvons même imaginer de prévoir des modules spécialement conçus pour les usagers du vélo. tout cela à un coût. À Montpellier, de lourds investissements ont été réalisés jusqu'en 2014. Il faut toutefois garder à l'esprit que la gratuité suppose, par définition, moins de recettes et un nécessaire redéploiement de certains personnels. Aujourd'hui, dans le cadre des mobilités du quotidien et de la lutte contre le réchauffement climatique, l'État est-il prêt à s'engager dans une politique globale en soutenant financièrement une métropole comme celle de Montpellier, si elle décidait la gratuité de ses transports et, naturellement, l'extension de son réseau ? Je pense notamment à une renégociation des encours de dette

La gratuité, comme l'ont montré les travaux du GART et de la mission dont on vient de parler, pose effectivement des questions de soutenabilité économique et doit être examinée au cas par cas pour en déterminer l'efficacité.

En effet, les recettes tarifaires des réseaux de ces métropoles, perçues auprès des usagers, représentent des sommes très importantes et couvrent une part significative des dépenses de fonctionnement. L'État n'a évidemment pas vocation à intervenir financièrement dans les politiques de transport, qui relèvent des collectivités locales. C'est pourquoi il convient que celles-ci considèrent avec la plus grande prudence les effets potentiels de la gratuité sur leurs ressources,

L'État souhaite continuer à favoriser le développement de projets structurants ; à ce titre, il continuera à soutenir de tels projets, avec un quatrième appel à projets en faveur des investissements en transports collectifs, lancé en 2020, la LOM ayant prévu des crédits à cette

mais à quel prix ? Les interventions d'aujourd'hui sont la preuve que le sujet de la gratuité des transports collectifs passionne et continuera sans aucun doute à faire parler de lui, surtout en cette période préélectorale. Je tiens à remercier tout d'abord les administrateurs, le rapporteur et l'ensemble des groupes politiques qui ont participé, de manière constructive, aux travaux de la mission d'information. Nous sommes parvenus à atteindre un équilibre qui, je dois l'avouer, n'a pas été facile à trouver. Le premier projet de rapport n'avait d'ailleurs été ni adopté ni rejeté, et nous avions choisi,

l'été. À la lumière des débats d'aujourd'hui, que faut-il retenir de la gratuité des transports collectifs ? D'abord, comme je le disais, c'est un sujet qui passionne, et pour cause

dès que nous tentons une réflexion un peu approfondie sur la question, il est indéniable que la gratuité ne saurait être présentée comme une réponse miracle adaptée à toutes les situations. Je reste personnellement convaincue que la gratuité, la gratuité totale, ne reste possible que dans certaines situations très spécifiques, dans lesquelles deux conditions sont réunies.

un financement qui repose essentiellement sur le versement transport. Dans ces cas très précis, seule la gratuité totale des transports collectifs peut servir, comme on l'a vu à Dunkerque, à renforcer l'attractivité du centre-ville ou encore à optimiser le service existant. J'avoue être beaucoup plus circonspecte, en revanche, sur les autres vertus que certains prêtent par ailleurs aux transports gratuits. Allez donc expliquer aux usagers du métro parisien, serrés à quatre par mètre carré aux heures de pointe, qu'il constitue un « lieu de vie » : succès garanti En outre, dans la très grande majorité des cas, la gratuité des transports collectifs reste une équation financière impossible à tenir pour les AOM en l'état actuel des financements, puisqu'elle implique à la fois la perte de recettes liées à la billettique, mais aussi une hausse des dépenses dues à l'augmentation de la fréquentation.

Plus encore, la question de la gratuité des transports collectifs, si elle reste une idée séduisante au premier abord, porte en elle le risque- cela a été dit -d'accroître les inégalités entre les zones urbaines, d'une part, qui disposent de réseaux de transports collectifs, et les zones rurales et périurbaines, d'autre part, où ils font souvent défaut. Comment justifier la gratuité des transports pour certains, alors qu'un grand nombre de nos concitoyens sont confrontés à d'importantes difficultés de mobilité dans de très nombreux territoires ? Je pense donc que la priorité doit rester le développement de l'offre de transport pour l'ensemble de nos territoires, et ce avant toute autre chose. Il y va de l'équité entre tous les Français. Les différentes auditions que nous avons menées dans le cadre de cette mission m'ont davantage convaincue de l'intérêt de développer une tarification équitable et lisible, une tarification solidaire pour les usagers, que l'on appelle communément la gratuité partielle. C'est la raison pour laquelle la mission a proposé la création d'un observatoire de la tarification des transports, qui permettrait aux AOM envisageant cette gratuité, qu'elle soit partielle ou totale, de disposer d'un outil spécifique. J'ai d'ailleurs demandé à monsieur le secrétaire

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en conclusion de cette mission, je crois pouvoir dire que la gratuité totale des transports collectifs ne constitue ni une bonne ni une mauvaise idée, mais un outil à disposition des collectivités pour contribuer, par exemple, à la revitalisation d'un centre-ville ou à la création d'un aménagement urbain qui laisse moins de place à la voiture. Il faut conclure, ma chère collègue. Fondamentalement, à travers cette question, c'est celle de l'inégalité territoriale qui est posée.

avons terminé avec le débat sur le thème : « Bilan et perspectives de la compétence " Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations " des inondations " . » Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, deux ans après son entrée en vigueur, il était important que nous ayons ce débat sur la mise en oeuvre de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Si nombreux étaient les élus réticents devant cette mesure, je pense aujourd'hui que c'était un mal nécessaire. Il nous fallait une gestion coordonnée de nos politiques en matière de milieu aquatique et de gestion des inondations.

À cela, s'ajoutait une absence totale de ressources humaines spécialisées sur ces questions. Ce sont aussi des questions de responsabilités qui ont présidé à la création de cette compétence. La recherche permanente par nos concitoyens de responsables nous a très certainement poussés à nous adapter. Les événements climatiques que nous avons connus dans les années 2010, comme la tempête Xynthia où les inondations dans de nombreux départements, sont venus étayer de manière parfois funeste ce constat. En attribuant cette compétence au bloc communal, le législateur de l'époque a assuré le lien essentiel entre politique d'urbanisme, gestion de l'eau, prévention des inondations, pouvoirs de police du maire et surtout proximité, qui sont déterminants en matière de Gemapi. Il est également venu poser l'obligation, pour les élus de chaque territoire, de définir en fonction de leurs spécificités la stratégie et les moyens à mettre en oeuvre pour l'amélioration des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Le texte tel qu'il avait été adopté comportait néanmoins quelques failles qui ne permettaient pas une mise en oeuvre harmonieuse et sereine de cette compétence. À ce titre, le travail effectué lors de l'examen de la loi portant votre nom, monsieur le ministre, loi qui est venue intégrer la « sécabilité », a permis le passage d'une compétence exclusive à un « chef de filât » et a autorisé les départements à continuer d'agir dans ces domaines, a été plus que bienvenu. Aujourd'hui, après presque deux ans de fonctionnement, où en sommes-nous ? S'il nous a fallu attendre longtemps la publication du rapport sur la mise en oeuvre de cette compétence, les remontées du terrain nous ont permis de nous faire un premier avis. d'abord, je dirai que la prise effective de compétence varie selon les territoires. La carte intercommunale, la perception des risques d'inondation, l'éventuel risque de submersion et les moyens financiers ont plus ou moins précipité la prise de compétence Gemapi. Et pour cause ! Pour nombre d'élus, la création de cette compétence est apparue comme un transfert de charges de l'État. Force est de constater qu'il n'a pas été accompagné des transferts financiers équivalents et nécessaires. Si vous demandez aujourd'hui à un élu quelle est sa principale préoccupation concernant la Gemapi, il vous répondra sans hésiter : le financement ! D'abord, parce que l'instauration de la taxe Gemapi est aujourd'hui laborieuse, seulement un tiers des Français la paye ensuite, parce que cette taxe dépend en partie d'une taxe d'habitation dont la compensation est actuellement encore hasardeuse ; enfin, parce qu'elle ne rapporte pas suffisamment. Qui peut penser que les 145 millions d'euros récoltés l'année dernière sur l'ensemble du territoire permettront de financer les ouvrages ?

Je le dis avec d'autant plus de liberté que ma collectivité fut l'une des premières à mettre en place la Gemapi. Dès 2017, au sein du Pays de Lourdes et des vallées des Gaves, que je présidais, nous anticipions cette prise de compétence pour permettre une gouvernance commune de ces enjeux à l'échelle du bassin versant du gave de Pau amont. Cette prise de compétence ne s'est pas faite sans conséquence puisque désormais c'est près de 1 million d'euros de budget qui sont destinés à la Gemapi sur ce périmètre. Or, même si nous étions précurseurs, de nombreuses questions restent aujourd'hui sans réponses et beaucoup d'élus ont l'impression d'être au milieu du gué, en termes de caractérisation de la compétence. Dans une question de décembre 2018, j'interrogeais par ailleurs Mme la ministre Jacqueline Gourault sur ce sujet, notamment sur la qualification de l'urgence. Lorsque surgit un événement climatique entraînant des crues et des débordements de cours d'eau, il est souvent difficile de dissocier, d'une part, la protection des ouvrages réalisés ou non par l'établissement public de coopération intercommunale n'étant pas classés en tant que systèmes d'endiguement et, d'autre part, la protection des enjeux, de la population et des biens, prérogatives dévolues au maire. D'ailleurs, il arrive bien souvent que les techniciens des entités chargées de la Gemapi viennent en appui pour réaliser des travaux afin d'éviter les inondations dans les zones habitées, mais aussi pour protéger les ouvrages dont la collectivité compétente pour la Gemapi a la charge contre les inondations. preuve que, si la définition de l'urgence est à établir, celle de l'intérêt général l'est tout autant. Ce constat soulève différentes interrogations. Tout d'abord, les maires peuvent-ils agir sur les ouvrages dont les EPCI ont la charge afin de prévenir d'éventuels dégâts dans le cadre de leurs pouvoirs de police en termes de prévention des inondations Cette question de coordination dans la décision se pose également pour la gestion des systèmes d'endiguement. On note d'ailleurs, pour ces derniers, que l'État se fait aujourd'hui beaucoup plus regardant sur l'entretien de ces digues depuis le transfert aux collectivités Il va donc falloir aller plus loin dans l'information des élus des autorités « gemapiennes » sur l'avancement de la mise en conformité des systèmes d'endiguement qui les concernent, avec une véritable programmation concertée des travaux pour aboutir à une cohérence entre les systèmes proposés et les attentes des collectivités. Même avec davantage de proximité, le financement de ces ouvrages restera incertain ! Les 15 millions annuels promis par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs pour les digues sont insuffisants. Certes, monsieur le ministre, vous allez me dire que la somme a été déplafonnée, mais ce n'est qu'une réponse partielle aux EPCI concernés. Une meilleure acceptation passera sans doute par une clarification des compétences en s'appuyant sur les piliers de l'organisation du bassin que sont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, pour le volet aquatique, les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI), concernant les inondations, et par une garantie des financements sur les programmes pluriannuels cadres comme les contrats de rivières ou les programmes d'actions de prévention des inondations. tels que ceux que je viens d'évoquer ne manquent pas par leur nombre ni par leur efficacité, leur mise en oeuvre est souvent laborieuse du fait des contraintes environnementales parfois incompatibles avec les soucis de prévention. Je pense sincèrement que le salut de la Gemapi passera par une sanctuarisation des budgets des agences de l'eau et par une réorientation du fonds Barnier, préconisée par le récent rapport de nos collègues Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart. Cette réorientation est une évidence lorsque l'on sait que, pour 1 euro de dépense en prévention, 7 euros sont économisés en réparation ! Monsieur le ministre, j'espère que vous aurez à coeur de répondre à nos interrogations qui sont nombreuses, notamment sur la gestion des dispositifs de défense contre la mer, la gestion des grands fleuves, mais aussi l'exercice de la Gemapi outre-mer. Mes chers collègues, j'espère que vous aurez autant d'intérêt que moi à débattre sur ce sujet ô combien important pour nos élus et pour nos concitoyens. La parole

La gestion des cours d'eau et celle du risque d'inondation sont liées. Elles nous obligent à penser de conserve la gestion des zones d'extension naturelle des crues et l'entretien des ouvrages de protection contre les inondations. Elle appelle à un défi technique, d'ingénierie et financier. C'est la raison pour laquelle la gestion de l'eau et la prévention des inondations devaient être rapprochées. Je suis donc heureux du débat que nous avons aujourd'hui sur ce sujet. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi Maptam, avait introduit par la voie d'un amendement sénatorial la compétence Gemapi, et en avait confié la gestion, à titre exclusif et obligatoire, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Elle partait du constat qu'il fallait préserver ce qui fonctionne. Ainsi la loi dispose désormais que les départements et les régions assurant une ou plusieurs des missions attachées à la compétence Gemapi peuvent poursuivre leurs engagements en la matière au-delà du du 1 janvier 2020- je pense, en particulier, à la prévention des inondations sur les côtes. Un certain nombre de départements étaient très engagés. Le texte tel qu'il était rédigé initialement ne leur permettait plus de poursuivre les actions menées. Par ailleurs, les cours d'eau, comme les crues, s'ordonnancent et se développent à une échelle qui leur est propre, celle des bassins versants. Elle échappe parfois à la logique des découpages administratifs. Dès lors, les limites administratives des collectivités territoriales ne sont pas adaptées à la disposition géographique des bassins. C'est la raison pour laquelle elles se sont réunies dans des syndicats mixtes, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (Épage) ou des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). C'est au sein de ces établissements qu'elles ont appris à travailler ensemble dans le cadre d'une coopération territoriale visant l'efficacité des politiques de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. La loi a donc introduit la possibilité de transférer ou de déléguer à un Épage ou à un EPTB une partie seulement des actions relevant de la Gemapi. De même, elle étend cette possibilité en cas de transfert de la compétence à un syndicat mixte de droit commun. Enfin, la loi étend désormais à la prévention des inondations les missions d'animation et de concertation, ainsi que l'assistance technique mise par les départements à la disposition des EPCI ne disposant pas des moyens techniques suffisants pour exercer leurs compétences. Nous avons souhaité en effet pouvoir conforter les collectivités et les aider à prévenir les inondations. C'est ainsi que le décret du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique est venu relever le plafond d'éligibilité des intercommunalités à l'assistance technique de 15 000 à 40 000 habitants, conformément à l'arbitrage rendu par le Premier ministre. Où en sommes-nous ? La compétence Gemapi, vous l'avez rappelé, madame la sénatrice, se structure progressivement et de manière différenciée : l'organisation de la compétence est aujourd'hui stabilisée ou en voie de l'être. Reconnaissons donc que la dynamique est enclenchée. Toutefois, nous constatons des disparités assez fortes entre territoires. En matière financière, l'article 56 de la loi Maptam du 27 janvier 2014 a instauré la faculté, pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, d'instituer la taxe Gemapi pour assurer l'exercice de leur compétence en la matière. Cette compétence est obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre depuis le 1 janvier 2018. La taxe Gemapi est un outil de financement puissant, clairement identifiable par la collectivité et par le redevable- le montant que ce dernier acquitte est explicitement mentionné dans son avis d'imposition qui contribue à la simplicité du financement de la compétence. La taxe Gemapi est affectée aux dépenses afférentes à la compétence et est plafonnée à 40 euros par habitant. J'entends ce que vous dites par ailleurs sur la question du financement, mais ce sont des moyens qui avaient été prévus par le législateur au Sénat. Une simple délibération de l'EPCI à fiscalité propre permet d'instituer la taxe, qui lui garantit une source de financement fiable dans la mesure où, d'une part, il adopte un produit et non un taux et où, d'autre part, la taxe est assise sur des impositions directes locales émises par voie de rôles et recouvrées par les services de l'État. La taxe Gemapi a connu une montée en puissance sensible depuis 2017.

En 2019, ce sont 556 EPCI à fiscalité propre qui ont adopté un produit de taxe Gemapi, soit 44 % du total. Ces EPCI regroupent une population de 32 millions d'habitants.

me semble primordial de faciliter et de simplifier la mise en oeuvre de la Gemapi en tenant compte des réalités locales et en faisant preuve de pragmatisme. Les collectivités locales se sont approprié de manières différentes ces compétences. D'abord, parce que certaines étaient directement et très régulièrement confrontées aux problèmes d'inondation.

de plus en plus fréquents et de plus en plus répartis sur le territoire amènent les collectivités à se saisir davantage de la question. Les services de l'État restent pleinement mobilisés pour accompagner les collectivités locales dans la prise de compétence Gemapi, en particulier dans les territoires où la gouvernance doit encore être confortée. Je pense, notamment, à la question des fleuves-

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons, la mise en place de la compétence Gemapi n'a pas été simple sur certains territoires. Je souhaite aujourd'hui porter à votre attention un exemple essentiel et spécifique : la précarisation de notre modèle de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Nous observons en effet un morcellement à la fois des entités et des méthodes, ce qui contribue à enrayer notre capacité à répondre aux attentes en termes de gestion de l'eau, et ce notamment en période d'urgence climatique. Deux points illustrent cette difficulté. Le premier se situe dans la fragilisation des équilibres et des principes de solidarité déjà existants. C'est notamment le cas de la Bresle, petit fleuve côtier qui sépare la Somme de la Seine-Maritime, où deux EPCI sur sept composant le bassin versant ne travaillent pas la main dans la main, que ce soit entre eux ou avec les autres collectivités territoriales. Cela nous amène au second point, qui concerne la clarification du périmètre des compétences, entre celles qui relèvent de la Gemapi et celles qui sont en dehors. Les problématiques liées au grand cycle de l'eau demandent une approche globale et intégrée. Plusieurs volets de la gestion de l'eau doivent être étudiés et envisagés : de nombreux pans sont à prendre en considération, passant tout autant par la qualité de l'eau que par sa quantité. Il faut également prendre en compte la biodiversité, vecteur essentiel de nos territoires, ou encore la préservation des ressources. Monsieur le ministre, à la lumière des deux points évoqués, pensez-vous utile d'organiser dans des délais raisonnables un débat approfondi sur la question de la gouvernance et du financement des politiques de l'eau à l'échelle des bassins versants ? je vous remercie d'inondations et de la Gemapi. Le comité de bassin constitue l'instance de concertation privilégiée pour tenir un débat sur la question de la gouvernance et du financement des politiques de l'eau à l'échelle des bassins versants. Regroupant différents acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine de l'eau-

des eaux pluviales et de ruissellement dont peu de collectivités souhaitent se saisir, faute de financement et de précisions apportées par la loi. Ces différents points devraient également être pris en compte dans le débat que vous nous avez proposé sur ces sujets.

de l'eau et de sa gestion, la mission du législateur n'est jamais simple. Comme c'est le cas pour la compétence « eau et assainissement », pour laquelle le débat n'est d'ailleurs toujours pas définitivement tranché, la compétence Gemapi aura eu un parcours législatif chaotique. Aujourd'hui, plusieurs acteurs participent à cette compétence : des EPCI, des syndicats mixtes, mais aussi les départements et les régions. Toutefois, cette pluralité, qu'avait tenté de supprimer la loi Maptam, n'est pas forcément la principale difficulté. Je souhaiterais insister sur les problèmes tenant à la mise en oeuvre de la Gemapi sur le littoral. Les acteurs se trouvent confrontés à un empilement de procédures administratives, financières et environnementales de toutes sortes. Surtout, on constate que, dans les faits, la décentralisation n'est pas allée à son terme. Sur le terrain, la multiplication des procédures, les éternels aller-retour avec l'administration centrale masquent alors l'arbitrage local. On se retrouve aujourd'hui face à une contradiction la lourdeur et la longueur des procédures s'opposent à l'urgence de protection des populations. Comment accélérer et simplifier les procédures ? En Vendée, je citerai notamment l'exemple du syndicat mixte du Marais poitevin bassin du Lay. Cet organisme chargé de la Gemapi a récupéré un ensemble d'ouvrages en ruine qui nécessiteraient trois ou quatre ans d'études préalables à leur remise en état. Il se retrouve alors dans une situation très délicate, puisqu'il est dorénavant seul responsable d'ouvrages, en l'occurrence des digues, pour lesquels la responsabilité est demeurée floue pendant près de soixante ans. C'est une situation souvent techniquement et financièrement intenable. moralement insupportable dans un département qui commémorera en février prochain les dix ans du drame de la tempête Xynthia. Enfin, je poserai une dernière question, plus concrète encore, monsieur le ministre : de quels moyens dispose l'autorité chargée de la Gemapi si elle souhaite faire une digue sur un tracé qui a été refusé

administratives complexes. Des simplifications importantes ont été apportées à la réglementation sur les ouvrages hydrauliques, notamment avec l'instauration de l'autorisation environnementale unique, qui permet d'accélérer un certain nombre de procédures. L'État est conscient de l'enjeu lié à la nécessité de réaliser des travaux rapidement, notamment à la suite d'une crue

Le rapport conclut qu'une modernisation de nos politiques de prévention et d'indemnisation est indispensable pour relever durablement le défi du changement climatique. Vous le voyez, monsieur le ministre, nous ne nous sommes pas uniquement focalisés sur les conséquences des catastrophes climatiques et donc sur le régime de catastrophe naturelle, intéressons à l'ensemble du phénomène, tout particulièrement à la prise en compte du risque, ce qui rejoint le débat que nous avons aujourd'hui sur l'initiative du groupe du Pour ces raisons, nous avons successivement proposé : de renforcer le rôle du conseil de gestion du fonds Barnier et de supprimer les sous-plafonds pour donner davantage de souplesse à sa gestion d'achever la politique d'élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) ; d'accélérer le traitement des demandes de labellisation des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) et de simplifier les procédures applicables aux actions réalisées dans ce cadre de créer des instruments juridiques adaptés aux territoires confrontés au recul du trait de côte ; enfin, de créer les conditions pour développer une culture du risque chez nos concitoyens. Pourquoi ce rappel ? Parce que le transport de la compétence Gemapi a profondément fait évoluer le rôle des élus, qui sont devenus acteurs de la prévention des risques, et ce alors même que la frontière entre ce qui relève de la Gemapi et ce qui n'en relève pas n'est pas claire, et que le modèle financier n'est pas réaliste. Ce n'est pas vous, monsieur le ministre, qui pouvez me contredire sur ce point. Surtout aussi, parce que le conseil ont été mandatés pour évaluer l'efficacité de la mise en oeuvre des PAPI et qu'ils sont, en ce moment même, en train d'examiner certaines des solutions que nous proposions dans nos travaux. Monsieur le ministre, ceux qui veulent faire

le régime des catastrophes naturelles, des réflexions sont en cours en lien avec les acteurs concernés pour améliorer l'efficacité du dispositif. Sur la prévention des risques, nous vous confirmons que le fonds Barnier est un levier essentiel du financement de la politique de prévention des inondations. Le plafonnement actuel de ce fonds n'obère pas son efficacité

Nous rejoignons aussi les recommandations du rapport visant à poursuivre et renforcer les actions de prévention : PPR, PAPI, développement d'une meilleure appréhension du risque, réduction de la vulnérabilité. de la vulnérabilité, je souligne que le taux d'aide aux propriétaires d'habitation par le fonds Barnier est désormais passé de 40 % à 80 % pour les PAPI. Il en sera de même pour les PPR dans les jours à venir. Je veux revenir à ce que vous avez dit sur le rôle des élus. Il est vrai que du fait de la prise de la compétence

un certain nombre d'élus nous ont fait part de leurs inquiétudes et du fait qu'ils souhaiteraient des évolutions dans le but d'optimiser et de mieux financer certaines opérations de lutte contre le ruissellement. En effet, dans certains territoires, c'est l'une des premières causes d'inondations. La taxe Gemapi définie à l'article 1530 du code général des impôts peut être mobilisée afin de permettre le financement des opérations de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, dès lors que ces opérations contribuent à réduire le risque d'inondation. Cela est d'ailleurs clarifié par la circulaire sur la mise en oeuvre de la loi Gemapi du 30 décembre 2017. Par exemple, les ouvrages hydrauliques conçus de manière à limiter les dommages des eaux de ruissellement peuvent être financés au titre de la compétence Gemapi. Toutefois, cette taxe ne peut pas être mobilisée pour réparer les dégâts causés par le ruissellement et l'érosion, et leur non-intégration au sein de la Gemapi empêche la mobilisation des fonds qui lui sont consacrés pour mener des actions de réparation, avec des coûts parfois très lourds pour les collectivités concernées, compte tenu de leur situation budgétaire. Par ailleurs, le rapport inscrit à l'article 7 de la loi, qui a été rendu en avril 2018, soulève la réflexion à mener pour mieux articuler le financement des opérations et équipements concourant à la prévention des inondations par la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement. Je souhaite donc connaître votre position, monsieur le ministre, sur l'éventuelle intégration de la lutte contre l'érosion et le ruissellement au sein de la compétence Gemapi, afin de permettre aux collectivités de mobiliser cette taxe pour ces opérations spécifiques, et sur les suites données aux recommandations de ce rapport. La parole

En effet, cette suppression laisse planer quelques incertitudes notoires quant à la composition de l'assiette de recettes de la compétence Gemapi, laquelle peine, chacun le sait, à s'adosser à un modèle économique stable. Je rappelle aussi, et vous l'avez confirmé précédemment, qu'il s'agit de plus de 150 millions

préconise de « fiabiliser l'assiette de la taxe, qui subira le contrecoup logique de la suppression de la taxe d'habitation ». En l'état, la suppression de cette taxe, sur laquelle est partiellement assise la Gemapi, emporte emporte le risque de déplacer la charge de son coût budgétaire des populations locales aux entités qui sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE), aurait pour effet d'instituer logiquement une asymétrie de traitement, dès lors que les propriétaires du bâti exposé tireront le principal bénéfice de la réduction de l'exposition au risque. Une attention particulière sera-t-elle portée

j'ai faite à M. Sueur. La refonte de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe d'habitation ne modifie aucunement la faculté laissée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre à fiscalité propre d'adopter un produit de la taxe Gemapi- je rappelle, en effet, que c'est sur un produit que l'on vote. Les communes et les EPCI à fiscalité propre continueront, dans les mêmes conditions, à pouvoir adopter annuellement un produit d'imposition affecté au dépensier à l'exercice de la compétence, et plafonné à 40 euros par habitant. L'article 5 du projet de loi de finances pour 2020, qui a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et sera débattu dans quelques jours au Sénat, est clair quant à l'assiette de la taxe Gemapi retenue après la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Contrairement à ce que vous dites, aucune incertitude notoire ne persiste. La refonte de la fiscalité locale modifie simplement les modalités de répartition du paiement de la taxe entre les redevables. En 2020, la taxe Gemapi sera répartie entre la taxe d'habitation, les taxes foncières et la CFE, mais le taux additionnel de répartition appliqué sur la taxe d'habitation sera identique à celui de 2019. Cela permet de garantir à 80 % des foyers fiscaux de ne payer aucune taxe d'habitation en 2020. Le produit supplémentaire éventuellement adopté par l'EPCI à fiscalité propre sera réparti sur les autres impositions. En 2021 et 2022, le montant de la taxe Gemapi réparti sur la taxe d'habitation sera diminué des dégrèvements accordés en 2020, pour éviter que les 20 % de foyers fiscaux restant temporairement assujettis à la taxe d'habitation ne soient confrontés à un ressaut de de fiscalité. À compter de 2023, le produit de la taxe Gemapi sera réparti sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la CFE. La part répartie sur la taxe foncière sur les propriétés bâties sera calculée sur la base du taux communal. Par construction, à produit de taxe Gemapi égal, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales entraînera un report de la répartition sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la CFE. Néanmoins, d'une part, ces modalités de répartition part, ces modalités de répartition ne modifient pas le pouvoir d'institution et de fixation du produit accordé aux communes et aux EPCI à fiscalité propre compétents ; d'autre part, la hausse de la pression fiscale sur les redevables a été analysée et n'est pas

usées par l'opposition des acteurs traditionnels de la prévention et par les querelles byzantines des théologiens du contrôle de légalité, à propos de « qui doit faire quoi » et de l'utilisation licite ou non de la taxe Gemapi. On leur doit la paralysie de nombreuses opérations visant à maîtriser le ruissellement,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi Maptam de 2014 a transféré aux EPCI à fiscalité propre la compétence Gemapi. La loi NOTRe de 2015 a fixé au 1 janvier 2018 la date d'effet de ce transfert. Enfin, la loi de 2017 a permis aux départements et aux régions de continuer d'exercer la compétence Gemapi. Ce qui était un assouplissement nécessaire pose aujourd'hui un problème d'exercice de la compétence au niveau local. Dans mon département de l'Aube, par exemple, le département assure maintenant seul la compétence, les syndicats de proximité ayant été supprimés. Leur fonction était pourtant essentielle. Nous avons besoin d'une approche qui soit la plus locale possible, pour bien gérer cette compétence, surtout compte tenu des effets du changement climatique. À ce jour, les maires constatent un retard dans la gestion de proximité et trouvent que le suivi n'est plus évident. La gestion des cours d'eau en milieu rural est devenue difficile. Monsieur le ministre, le rapport de novembre 2018 sur le bilan du transfert de la compétence constate que son accompagnement doit être renforcé. Qu'est-il donc prévu pour assurer l'exercice local de la compétence Gemapi dans les zones où le chef de filât est assuré par les régions et départements ?

Dans de nombreux territoires, les départements sont en effet des partenaires importants des politiques de l'eau. Ils interviennent notamment dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, apportant leur soutien financier ou une assistance technique pour certaines opérations d'investissement.

pour accompagner les collectivités dans la prise de compétence Gemapi. Des outils d'accompagnement sont d'ores et déjà disponibles. À titre d'exemple, au niveau national, des guides à destination des élus et des techniciens sont désormais disponibles. Un guide sous

Les élus locaux, malgré leur engagement, attendent que l'État donne une impulsion réelle pour la reconquête de la qualité des eaux. J'aimerais vous faire part de plusieurs observations d'élus chargés de l'eau dans mon département.

Le deuxième point est la clarification de la gouvernance locale en matière de grand cycle de l'eau, qui n'est pas toujours une réalité : entre les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage), les départements, les régions et les EPCI, on constate encore une trop grande dispersion des initiatives et une sédimentation des responsabilités. Il faut vraiment veiller à mettre en place des actions de simplification pour, au moins, déterminer quelle échelle demeure prescriptive sur les autres. Troisième observation : la compétence Gemapi, qui est

ne souhaitent pas mener d'actions concomitantes pour la gestion d'une rivière. C'est problématique pour l'amélioration du bon état écologique de certains cours d'eau. milieux aquatiques (GEMA) est fortement subventionnée par la région et l'agence de l'eau par le biais des contrats territoriaux milieux aquatiques. La prévention des inondations, en revanche, n'est pas subventionnée. L'État prévoit-il la mise en place d'aides au financement sur ce poste ?

EPTB couvrant les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, a lancé une étude d'opportunité de classement des systèmes d'endiguement. Les résultats et propositions de cette étude vous ont été transmis. Il en ressort que le système d'endiguement semble être un outil réglementaire inadapté. Les territoires ruraux, qui disposent de longs linéaires de digues protégeant l'habitat diffus contre les inondations, auront d'énormes difficultés financières à maintenir ces ouvrages classés, et ce malgré l'instauration de la taxe Gemapi. Cette ressource financière est par ailleurs remise en cause par la suppression de la taxe d'habitation. À titre d'exemple, la mise aux normes de la digue de la rive droite de l'Adour maritime, longue de 23 kilomètres, qui protège 350 personnes, est estimée à 33 millions d'euros., d'euros., certains ouvrages non classés ne peuvent pas non plus être abandonnés, en raison de la présence de population, d'activités économiques agricoles ou d'enjeux de préservation de sites protégés Natura 2000, comme les barthes de l'Adour. Dans cette perspective, la proposition du décret d'août 2019 consistant à supprimer le seuil plancher de 30 personnes pour le classement des ouvrages n'est pas une solution. Il expose les entités « gemapiennes » à une situation inextricable, compte tenu du faible nombre d'habitants, et alors que les EPCI n'ont déjà pas les moyens financiers de classer des ouvrages protégeant des populations importantes. Au-delà de cette impasse financière, cette proposition apparaît contraire à la compétence Gemapi, puisqu'elle est de nature à maintenir des contraintes au fonctionnement naturel des cours d'eau. Ma question portera donc sur trois points. Comment les entités « gemapiennes » vont-elles supporter le financement des ouvrages classés avec cet abaissement de seuil et la fragilisation de l'assiette de la taxe Gemapi ? Pouvez-vous clarifier le devenir des ouvrages non classés au regard de l'obligation de mise en transparence hydraulique issue du décret de 2019 ? Qui sera chargé de la réaliser ? En conséquence, ainsi que le président de l'Institution Adour vous l'a proposé, êtes-vous favorable à la création d'un nouvel outil administratif réglementaire, garantissant la sécurité publique, adapté aux territoires ruraux et qui serait assorti d'un dispositif d'accompagnement financier soutenable ?

Certains acteurs pensent que l'ancienne réglementation leur permettait de conserver les digues protégeant moins de 30 personnes sans être soumis à la réglementation. Or ce n'est pas le cas : la loi prévoit en effet que ces digues non intégrées à un système d'endiguement doivent être neutralisées, c'est-à-dire supprimées. L'ancienne réglementation aboutissait donc à supprimer automatiquement les digues protégeant moins de 30 personnes. La nouvelle réglementation permet de conserver ces digues si la collectivité le souhaite, pour répondre précisément à la question que vous avez posée. Mais cela n'est pas une obligation

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est désormais une habitude pour notre Haute Assemblée, je dirais même une figure imposée des débats sur les compétences des collectivités territoriales : je compte moi aussi vous parler d'eaux pluviales. Pourquoi évoquer ce sujet ? Cette question est-elle encore d'actualité avec la loi du 3 août 2018 ? Si oui, un débat sur la Gemapi est-il le bon véhicule ? le bon véhicule ? Cette question, en apparence simple, est le plus beau symbole du dédale technocratique dans lequel on plonge les élus locaux. En conséquence, la question « Qui s'occupe des eaux de pluie en France ? » nécessite davantage de développements que le code du travail suisse.

et le reste des eaux pluviales que l'on nomme « eaux de ruissellement ». S'agissant de la compétence « eaux pluviales urbaines », celle-ci est obligatoirement exercée à l'échelon intercommunal, sauf pour les communautés de communes depuis la loi précitée du 3 août 2018. S'agissant des eaux de ruissellement, il semble que nous soyons toujours en présence d'un angle mort. Cette compétence ne relève pas de la gestion des eaux pluviales urbaines ni de l'assainissement, et elle n'est que voisine de la Gemapi. Par défaut, la jurisprudence la classe avec la voirie. De fait, ni le rapport d'avril 2018 sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations ni le rapport de l'IGA et du CGEDD du 21 octobre dernier n'offrent de réponse claire. Alors, vers quelle formule nous dirigeons-nous Cette compétence « eaux de ruissellement » sera-t-elle un jour rattachée à la Gemapi ? Ou allons-nous assister, comme le propose le CGEDD,

vous l'avez rappelé, dans son rapport au Parlement prévu par les dispositions de l'article 7 de la loi du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la Gemapi, le Gouvernement a souligné la diversité des moyens techniques pouvant être mobilisés pour assurer une gestion efficiente des eaux pluviales. des eaux pluviales. Je rappellerai le schéma dans lequel nous évoluons. Pour les communautés urbaines et les métropoles, la loi rattache désormais explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence « assainissement

et de la prévention des inondations. Ainsi, il fallait concilier la clarification juridique de la répartition des compétences exercées par les collectivités territoriales et la souplesse utile à la mise en oeuvre de ces compétences. C'est bien l'objet des dispositifs qui ont été votés par les parlementaires. Dès lors, identifier spécifiquement la compétence « eaux pluviales urbaines » et la confier obligatoirement, à l'instar de l'assainissement, aux métropoles et aux communautés urbaines à compter du 1 janvier 2020 constitue une clarification institutionnelle. C'est aussi une simplification financière, car la gestion des eaux pluviales étant une compétence distincte, il n'est plus obligatoire de la financer par le budget de l'assainissement : il pourra être recouru au budget général, voire à la taxe Gemapi, si le traitement des eaux pluviales est lié, comme c'est parfois le cas, à la prévention des inondations par exemple. Cette compétence demeurera cependant facultative pour les communautés de communes. Il est ainsi laissé

le groupe socialiste et républicain ce que l'on peut tout à fait comprendre, votre gouvernement a institué un plafond de recettes à hauteur de 12,6 milliards d'euros. Avec ce plafond, les six agences se voient amputées de plus de 1 milliard d'euros par rapport au dixième programme. Cette situation induit mécaniquement la diminution et l'arrêt de certaines aides aux collectivités territoriales qui sont toujours nécessaires pour mener à bien les compétences « eau », dont la Gemapi. Pourtant, il est plus que jamais indispensable de donner aux agences de l'eau les moyens de faire face aux défis liés au réchauffement climatique et à la dégradation des milieux aquatiques, comme il est nécessaire de donner aux collectivités les moyens d'exercer leur compétence « eau « eau ». Monsieur le ministre, il faut revenir au principe selon lequel « l'eau paie l'eau ». La compétence Gemapi justifie que les agences de l'eau apportent leur aide aux établissements chargés, pour le compte des EPCI, de la gestion des bassins versants. Le lien est évident entre biodiversité, fût-elle cultivée, des bassins versants et qualité des milieux aquatiques, et donc de la ressource en eau. Les agences de l'eau sont les mieux placées pour faire le suivi et la synthèse de la relation entre l'eau et la biodiversité à l'échelle des bassins versants.

souligné l'importance de ces actions. Je rappelle qu'un « aqua prêt » de la Caisse des dépôts et consignations a été mis en place pour financer des actions. Près de 57 millions d'euros de prêts ont déjà été engagés au premier semestre de 2019. En ce qui concerne les

La loi de finances pour 2018 a mis en place un plafond mordant pour les redevances des agences de l'eau, vous l'avez rappelé. Le onzième programme d'intervention des agences prévoit cependant un accompagnement des actions de Gemapi, dès lors qu'elles sont corollaires aux actions de préservation des milieux aquatiques.

Lopez. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je viens d'un département fortement soumis aux caprices du temps, le Gard- vous pouvez l'entendre à mon accent ! -, dans lequel la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations fait presque l'objet d'une obsession collective, tant elle a pu impacter tragiquement le quotidien de ses habitants. Jugez plutôt : depuis la moitié du XIII siècle, le Gard a connu plus de 500 crues. L'équinoxe d'automne représente pour nous la période la plus critique. Vous comprendrez donc aisément qu'à cette période chaque grosse pluie soit attendue avec tant d'appréhension. Chacun a en effet en mémoire la terrible catastrophe du 3 octobre 1988

avec 22 morts, 299 communes du département sinistrées sur 353 et plus de 830 millions d'euros de dégâts. Face à ce constat, la nécessité de réduire durablement la vulnérabilité de notre territoire est apparue comme une évidence. Différents acteurs se sont donc attachés, avec plus ou moins de succès, à mener successivement des actions visant à réduire l'impact des inondations sur les personnes, les biens et les activités économiques, avec la création de syndicats départementaux, régionaux, puis interrégionaux, le déploiement de moyens pour l'endiguement et la création de bassins de rétention, pour en citer les principales. Pourtant, le principe de la protection contre les risques naturels n'a jamais été remis en cause et relève le plus souvent des habitants ou des propriétaires généralement regroupés en associations. L'aménagement du territoire, et particulièrement l'organisation des zones urbanisées, doit aujourd'hui intégrer, outre la satisfaction des besoins liés au logement et aux activités économiques, les atteintes liées à la sécurité des personnes et des biens et celles liées à la qualité de vie et à l'environnement. La directive-cadre sur l'eau et la directive Inondations ont fixé un cadre et des objectifs ambitieux en matière de gestion équilibrée de la ressource en eau. La mise en place de la compétence Gemapi répondait ainsi opportunément à un besoin de cohérence de l'action publique, de replacement de la gestion des cours d'eau au sein des réflexions sur l'aménagement du territoire, de recentralisation des différents acteurs pour une meilleure efficacité. Force est ainsi de reconnaître, à deux mois à peine de la date butoir de la mise en place obligatoire de la compétence Gemapi, qu'il subsiste encore de véritables questions.

le 27 janvier prochain, cela fera six ans que le processus de transfert de la compétence Gemapi a été engagé. Six ans plus tard, la discussion autour de l'exercice de cette compétence n'est pas close. Ce débat de contrôle demandé par nos collègues du groupe du RDSE en est une preuve flagrante. Au contraire, avec la loi dite Fesneau, puis avec la loi dite Ferrand, et enfin avec le projet de loi Engagement et proximité, nous assistons à une inflation législative sur le thème, preuve que ce transfert de compétence ne s'est pas déroulé dans les conditions que les élus appelaient de leurs voeux. Car, contrairement à ce que certains imaginent, si les élus n'ont pas été enthousiastes à l'idée de se voir confier une compétence qui relève bien souvent de la sécurité publique, et donc du pouvoir régalien, ils ont assumé leurs responsabilités. Mais puisque cette compétence a été transférée, et certains arguments en faveur de ce transfert sont pertinents, les législateurs que nous sommes demandent, dans le cadre du pouvoir de contrôle qui est le leur, que ce transfert de compétence soit accompagné des moyens nécessaires à son exercice. Or les interventions d'aujourd'hui, quelles que soient les étiquettes partisanes, montrent que tel n'est pas le cas. Ma question va donc relayer l'intervention de mes collègues, et notamment celle de Patricia Morhet-Richaud, qui évoquait la sous-consommation des crédits européens. Personne ici ne souhaite que la taxe Gemapi ou les redevances des agences de l'eau deviennent les seules variables d'ajustement d'une compétence trop lourde à porter. ministre, souhaitez-vous, comme l'évoque le rapport de l'IGA et du CGEDD d'octobre dernier, que les aides européennes puissent être fléchées vers des programmes stratégiques sur l'eau ? Surtout, êtes-vous en mesure de nous garantir que la future période de programmation 2021-2027 donnera plus de place aux projets qui correspondent aux axes de prévention des risques et de protection de l'environnement ? La parole

Elle transfère de façon exclusive et obligatoire la compétence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en associant deux volets aux problématiques bien différentes : la gestion des milieux aquatiques d'une part, la prévention des inondations d'autre part. La loi fait référence à quatre items : l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. Aux différentes actions relevant de la Gemapi, différentes solidarités sont associées : la solidarité interne aux EPCI, la solidarité de bassin et la solidarité nationale.

Parmi les quatre items du code de l'environnement, il est également difficile de distinguer ce qui relève de la gestion des milieux aquatiques, du « GEMA », et ce qui relève de la prévention des inondations, du «

l'État a imposé aux EPCI la compétence Gemapi, mais il a une importante responsabilité à assumer, stratégique et opérationnelle certes, mais aussi financière. À fiscalité constante, comment clarifier la compétence Gemapi sans transférer toute la responsabilité de la politique de l'eau aux communes et intercommunalités, dont beaucoup risquent de se retrouver dans une situation critique face à la multiplication des événements climatiques extraordinaires ? La parole

Madame la présidente, mes chers collègues, le moment est venu pour moi de remercier M. le ministre d'avoir bien voulu se prêter à cet échange. Je remercie bien évidemment les sénatrices et les sénateurs qui nous ont fait l'honneur de leur participation de s'être exprimés librement sur ce sujet d'ampleur, enrichi des situations rencontrées localement, mais aussi les nombreux élus qui ont assisté à ce débat. Le 21 octobre dernier, paraissait donc, après plusieurs mois d'attente, le rapport de la mission du CGEDD sur l'évaluation des conséquences de la mise en oeuvre des compétences dans le domaine de la Gemapi. Certaines préconisations d'évolution ont pu recueillir pleinement notre attention et ont été citées dans le débat, comme le dialogue renforcé entre l'État et les EPCI qui doit nécessairement s'établir concernant le transfert de la gestion des digues. Il plaît au Sénat de prendre appui sur ces travaux de fond pour dresser le bilan des évolutions des politiques publiques. Deux ans après l'adoption de la loi Gemapi et du transfert de la compétence, le présent débat n'a eu d'autre ambition que de poser les termes généraux d'un bilan, qui devra nécessairement être prolongé et entrer en résonance lors de l'examen du projet de loi Décentralisation, différenciation et déconcentration. Dans cet hémicycle, un constat commun est ressorti faciliter la mise en oeuvre de la Gemapi appelle nécessairement un réexamen du positionnement de l'État pour la prise en compte de la diversité des situations territoriales. En préambule, j'évoquerai la nécessité de mettre en place un suivi harmonisé de la Gemapi qui fait encore défaut, grâce à une évaluation régulière tant à l'échelon national

La mobilisation de la taxe Gemapi pour certaines opérations de lutte contre le ruissellement constitue une piste intéressante à développer. Concernant le modèle économique de la Gemapi, plusieurs points ont été soulevés le souhait de voir se pérenniser les financements de l'État, mais également des questionnements sur les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation sur la Gemapi. Vous y avez répondu, monsieur le ministre. Vous l'avez souligné dans votre discours, des disparités assez fortes entre territoires existent dans la structuration de la compétence Gemapi. Par cohérence, il est clairement apparu dans le débat qu'un accompagnement accru de l'État est attendu en fonction de la diversité des territoires. Dans les outre-mer, l'appropriation pleine et entière par les EPCI de cette compétence doit être un chantier mené par l'État. Les assises des outre-mer de 2018 avaient mis en lumière la nécessité de consolider les ressources en matière d'ingénierie et d'animer des réseaux de professionnel avec le Centre Dans les territoires concernés par le transfert, en 2024, des digues domaniales aux EPCI, les objectifs et les moyens financiers et humains pour la remise en état de ces digues posent légitimement question. D'autant plus qu'il y aura bien, à ce moment-là, transfert aux collectivités territoriales d'une nouvelle charge, considérable, sans compensation. Je mesure donc l'inquiétude des élus, qui devront composer avec des finances contraintes et qui savent le coût de ces ouvrages concourant à la Gemapi et de leur remise en état. Enfin, dans les zones littorales, qui peuvent être menacées par l'érosion ou la submersion marine, le périmètre de l'EPCI apparaît largement inadapté, qu'il s'agisse du niveau du périmètre de gestion ou des ressources financières mobilisables. En conclusion, je vous remercie au nom du groupe du RDSE d'avoir contribué à enrichir ce débat sur le bilan de la compétence Gemapi que nous aurons bien évidemment l'occasion de poursuivre- je l'espère en tout cas -lors de l'examen du projet de loi Décentralisation, différenciation et déconcentration. Nous en des inondations " . » J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.